La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public solennel sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale

le projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, puisque c'est désormais son nom, a fait l'objet ici, au Sénat, de modifications qui ne sont pas seulement cosmétiques. Je tiens à saluer le travail de la commission spéciale, qui a fait oeuvre de simplification, de précision et d'amélioration du texte issu de l'Assemblée Je retiendrai trois avancées majeures permises par le Sénat sur ce texte, qui illustrent, à mon sens, l'évolution du rôle de notre assemblée dans l'équilibre institutionnel de notre Le premier rôle, le rôle traditionnel du « grand conseil des communes de France », comme disait Gambetta, c'est bien sûr la défense des droits des collectivités dans la République. Notre assemblée a ainsi permis d'inscrire dans la loi l'extension du bénéfice du droit à l'erreur aux collectivités territoriales dans leurs relations avec les administrations de l'État. Cette mesure doit encourager un climat de confiance entre les différents degrés d'administration de la République, alors qu'aujourd'hui la défiance, ou disons la distance, est souvent la règle. La grande réforme de la fiscalité locale annoncée par le Gouvernement devra être empreinte de cet esprit, tant le respect et la confiance entre les acteurs locaux et centraux sont nécessaires à l'unité de la Nation et au bon fonctionnement de la République. Le Sénat est également un défenseur traditionnel de la ruralité française. Au moment où il est de bon ton d'instrumentaliser l'opposition entre les villes et les campagnes, il est indispensable que notre assemblée continue de créer des ponts, des liens, et d'apporter des solutions concrètes à nos concitoyens. Par exemple, l'amendement visant à reporter l'obligation de télédéclaration et de télépaiement pour les contribuables vivant dans les zones blanches est une mesure de justice à l'égard des territoires les plus reculés, qui ne doivent pas être des territoires oubliés. La suppression de l'article 34, défendue par les élus de notre groupe et d'autres, avait également pour objet de soutenir les petits producteurs d'énergie renouvelable en autoconsommation, souvent établis dans les zones rurales. Je me réjouis qu'elle ait été adoptée. L'écologie ne doit pas être réservée à ceux qui en ont les moyens. Au contraire, elle doit devenir un mode de vie concret et abordable pour tous les Français, où qu'ils soient, et sans logique punitive. Les membres de notre groupe défendent ainsi une croissance durable, inclusive et responsable, qui ne laisse personne sur le bord de la route. Le Sénat a, enfin, développé une expertise qui est la conséquence logique de ses rôles traditionnels que je viens de rappeler. Je veux parler de la défense des intérêts des très petites entreprises, les TPE, et des petites et moyennes entreprises, les PME, qui font la richesse de notre économie et le dynamisme de nos campagnes. Nous l'avons montré lors des discussions consacrées au dernier projet de loi de finances. Nous l'avons montré à nouveau lors de l'examen de ce texte, en prenant par exemple en compte la spécificité des plus petites entreprises en matière de prélèvement à la source ou en limitant la durée cumulée des contrôles administratifs

Notre collègue Emmanuel Capus a ainsi défendu l'extension aux entreprises de moins de vingt salariés des mesures dérogatoires prévues par le code de la sécurité sociale en matière de contrôle, pour alléger les normes pesant sur les petites entreprises. Nous avons également souhaité assouplir le délai de remise des pièces dans le cadre d'un examen de comptabilité, à la demande du contribuable et après validation par l'administration, pour les plus petites entreprises.

Nous sommes convaincus qu'un redressement durable de l'économie nationale passera par des mesures ciblées en faveur des PME. En Allemagne, ce sont les PME qui exportent, ce sont elles qui créent de l'emploi, ce sont elles qui innovent. En France aussi, mais elles subissent davantage de difficultés, car ce sont elles qui ont peur d'embaucher un salarié supplémentaire, ce sont elles qui n'ont pas les moyens de traiter la multiplicité et la complexité des normes, ce sont elles qui manquent d'accompagnement à l'export. Le changement de culture administrative, qui est l'ambition de ce projet de loi, devra donc s'adresser aussi à ces désabusés de l'administration que sont les dirigeants de TPE et PME. Collectivités contre État, villes contre campagnes, grandes entreprises contre petites entreprises : notre assemblée a pour vocation de réconcilier ces intérêts particuliers pour contribuer à la formation de l'intérêt général. Pourquoi opposer les uns aux autres, le Français des villes et le Français des champs, le fonctionnaire et le chef d'entreprise, le maire et le préfet ? notre groupe prennent acte de la volonté du Gouvernement et du Président de la République de restaurer la confiance entre l'administration et ses usagers. Nous les y aiderons en votant ce texte, avec les modifications, souvent bonnes, et parfois moins bonnes, qu'a apportées le Sénat. Nous souhaitons que la confiance, et non la méfiance, soit au coeur de l'ensemble des politiques publiques. C'est le sens de la démarche de mon groupe, ici au Sénat, de soutenir toutes les mesures qui vont dans le sens de l'intérêt général et de s'opposer aux divisions stériles et parfois artificielles. Enfin, en retenant, au sein de notre assemblée, les termes « relation de confiance » pour définir l'objectif de ce projet de loi, que voulions-nous dire ? Je crois qu'en un sens nous avons voulu exprimer une aspiration que les anciens appelaient « concorde », que les Constituants de 1848 appelaient « fraternité », valeur inscrite depuis dans notre devise nationale. Quel que soit son nom, confiance, concorde ou fraternité, cette idée d'unité a toujours présidé à la prospérité de la France. Ce texte, modeste en vérité, ne restaurera pas à lui seul la confiance dans la société française, qui est un édifice bien plus vaste. Mais, s'il peut constituer une petite pierre de cet édifice d'intérêt général, les membres du groupe Les Indépendants- République et Territoires le soutiendront ! La parole

Or nous sommes tous, dans cette assemblée, des sénateurs égaux les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas de raison pour que les sénateurs faisant partie d'un groupe

qui modifie dans une certaine mesure les rapports entre l'État et certaines religions. À mon sens, il n'est pas acceptable de voter un tel article à la sauvette, sans qu'il y ait un véritable débat. Stop ! La moindre des choses aurait été de consacrer

pour avoir su conduire cette expérience de façon subtile, et démontrer ainsi toute la pertinence de ce format -, madame, monsieur les rapporteurs de la commission spéciale, mes chers collègues, certains connaissent ici mon attachement particulier à Georges Clemenceau. Je ferai donc référence, aujourd'hui, à sa circulaire du 13 décembre 1917 intitulée « Réforme des méthodes de travail »,

Aujourd'hui, effectivement, l'heure présente exige davantage d'efficacité, d'adaptabilité, notamment digitale, et de bienveillance de la part de notre administration envers l'ensemble des usagers, qu'ils soient citoyens, entreprises ou collectivités locales- dans le présent texte par la commission spéciale du Sénat. Mais, dans les relations de l'administration avec son public, comment mener cette « chasse obstinée à tous les temps morts qui ralentissent encore la machine administrative » ? Georges Clemenceau nous donne la réponse c'est par la conversation, car « c'est affaire aux deux interlocuteurs de prendre leurs responsabilités et aussi leurs sûretés » : il ne faut recourir aux pièces écrites « qu'au moment voulu, c'est-à-dire lorsque l'affaire est [ ...] tout au moins dégrossie par la conversation La conversation ou, pour le dire de façon plus moderne, le dialogue doit se concevoir aujourd'hui comme un élément clef d'une relation entre l'administration et les administrés. C'est pourquoi les membres du groupe du RDSE approuvent l'objectif du Gouvernement d'encourager la constitution d'une administration plus à l'écoute et plus accessible pour accompagner ses usagers. il était tout aussi fondamental de maintenir les fonctions de contrôle et de prescription de l'administration. Les membres de notre groupe se félicitent donc que le Gouvernement partage leur avis quant à l'opportunité de supprimer un cadre « contractuel » à l'article 7. L'introduction de mesures telles que la mise en place d'un référent unique, la fin des appels surtaxés et l'introduction du rescrit sont encore, pour nous, autant d'éléments propices à la « conversation » entre l'administration et ses usagers. Dans sa circulaire, Clemenceau insistait sur le fait que chacun des acteurs devait prendre « ses responsabilités et ses sûretés ». Les élus de notre groupe accueillent donc favorablement l'introduction d'un « droit à la régularisation » pour les usagers dans leurs démarches administratives.

ce qui concerne les sûretés, le projet de loi consacre un « droit au contrôle », afin de permettre au public de faire examiner par l'administration la conformité de ses démarches. Enfin, ce texte responsabilise notre administration en dotant les usagers d'un « droit à l'opposabilité » quant aux conclusions des contrôles administratifs. Si ce projet de loi semble vouloir mettre en oeuvre un dialogue fluidifié et bienveillant entre l'administration et son public, nous regrettons que toute la place n'ait pas été laissée au Parlement pour converser sur ce texte. En effet, les élus du groupe du RDSE déplorent un recours excessif aux ordonnances. Avec douze demandes d'habilitation, certains sujets cruciaux, comme l'avenir des chambres d'agriculture, n'ont pas eu le débat qu'ils méritaient. Après le recours au vote bloqué sur la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricole, nous aurions souhaité avoir un débat conclusif quant au transfert de compétences entre les chambres d'agriculture départementales et régionales. Enfin, comme vous l'avez remarqué, au cours de l'examen de ce texte, les élus du groupe du RDSE se sont attachés à défendre avec force leurs convictions, avec leurs amendements relatifs à la loi du 9 décembre 1905. Oui ! Oui, la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est bien modifiée à deux reprises dans ce texte, par l'article 25, le code monétaire et financier, et par l'article 38 de ce projet de loi, qui vient modifier directement l'article 19 de la loi de 1905. Cette loi de 1905 fait de la France un État laïque et, par sagesse, rejette toute demande d'avantages spécifiques aux associations cultuelles. Les modifications introduites sont donc tout sauf anodines, dès lors que l'on touche au coeur des principes à valeur constitutionnelle de notre République. De surcroît, elles introduisent des inégalités de traitement entre les associations cultuelles et non cultuelles. La première mesure permet aux associations cultuelles de tirer profit d'immeubles de rapport pour aller au-delà de leur seule subsistance, alors que des associations loi de 1901 ne bénéficient pas d'autant de largesses. mesure permet aux associations cultuelles de ne plus être soumises aux mêmes obligations que les autres associations, pour ce qui concerne la notion de représentant d'intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP. Monsieur le secrétaire vous nous avez assurés, en séance, de votre « attachement viscéral voire radical à la laïcité »,, les élus du RDSE déplorent aujourd'hui l'ouverture d'une brèche importante dans la loi de séparation des Églises et de l'État. Ah, maintenant ça suffit ! ... je citerai encore quelques passages de sa circulaire. « Il faut traiter les affaires en hommes d'affaires : donc aller vite. » « On ne doit pas tolérer qu'un dossier soit transmis de porte en porte " pour attributions " [ ...] alors qu'une entente téléphonique lui eût assuré d'emblée sa légitime destination. » Il est inadmissible [ ...] de voir deux bureaux entreprendre un long échange de correspondance pour un renseignement qu'aurait fourni une conversation de deux minutes. » « Ces habitudes prises, on constatera que [ ...] 80 % des affaires peuvent être étudiées et résolues très rapidement. » Mes chers

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, nous procéderons tout à l'heure au vote solennel du projet de loi nouvellement dénommé au Sénat « renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public Je pense que chacun, dans cet hémicycle, s'accorde sur la volonté de placer la confiance au coeur des rapports entre l'administration et les Français. Oui ! Au sein du texte déposé devant le Parlement, deux mesures devaient tout particulièrement y contribuer la généralisation d'un droit à l'erreur et la création d'un droit au contrôle. Le droit à l'erreur, mesure centrale de ce texte de loi, au point de lui avoir donné son premier intitulé, permettra à l'administré de ne pas souffrir des conséquences d'une erreur commise bonne foi et pour la première fois. Ce nouveau droit, déjà mis en oeuvre par l'administration fiscale, viendra s'appliquer à de nombreux domaines du quotidien des citoyens, apaisant et facilitant ainsi leurs rapports avec l'administration.

permettant d'informer, d'orienter et de conseiller le public n'exclut pas le contrôle. L'extension du rescrit administratif, la création de certificats d'information et surtout la consécration d'un droit au contrôle découlent de cet impératif. Ces mesures servent toutes à fixer les bornes claires et nécessaires de la confiance. Mais, dans les faits, l'essentiel de nos débats n'a pas porté sur ces nouveaux droits et sur leur application. En effet, ceux-ci ne représentent qu'un quart environ du texte qui nous a été soumis. Le reste est constitué d'un ensemble de mesures couvrant des domaines très variés. Elles visent à simplifier et à modifier le droit existant, mais aussi à accompagner la dématérialisation de l'administration, ou encore, et surtout, à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance. C'est la raison pour laquelle ce texte a été qualifié de « fourre-tout » assemblant des mesures hétéroclites placées à la remorque de deux droits innovants. C'est aussi la raison de nos critiques portant sur la forme et sur la méthode. Le Président de la République lui-même affirmait, lors de son discours devant le Congrès, en juillet 2017, qu'il fallait « une activité parlementaire revivifiée par un cap clair [et] des débats mieux construits. texte, convenons-en, n'illustre pas ces beaux principes. Était-il nécessaire d'y inclure tant de recours à la législation par ordonnance ? Alors que souffle le vent de l'antiparlementarisme,

Pourquoi, d'ailleurs, diluer autant l'impact et la clarté de ce projet de loi ? Était-il nécessaire, pour légiférer sur la confiance, d'inclure des dispositions sur la géothermie, ... Oui ! ... sur les modalités de recouvrement des indus des prestations sociales, ou encore sur les modes de garde de la petite enfance ? La clarté et l'intelligibilité de la norme, qui sont des objectifs à valeur constitutionnelle, en souffrent grandement ! Et pourquoi attendre le dernier moment pour déposer certains amendements sur des sujets importants, ... Eh oui ! ... qu'il s'agisse d'engager une nouvelle expérimentation- la dix-huitième, excusez du peu -ou de revenir sur la décision d'attribution d'appels d'offres pour la réalisation de champs éoliens en mer ? Exactement ! Ce n'est manifestement pas là une marque de confiance. C'est un manque de respect et une très mauvaise manière faite au Sénat, que nous ne pouvons accepter. en oeuvre la confiance, c'est savoir laisser au Parlement la possibilité et le temps de préparer autant que de discuter la loi. C'est son rôle.

Contourner le Parlement pour mieux le contraindre, cela ne me semble pas porter le symbole d'un monde nouveau ... C'est vrai ! En voulant faire voter à la hâte des mesures aussi nombreuses qu'hétéroclites, on retire au Parlement la possibilité d'avoir un débat clair et mieux construit sur chacune d'entre elles. ne méritent-elles pas leur propre texte, qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur, des énergies renouvelables, des agences de notation ou de bien d'autres sujets encore ? Le chef de l'État n'était-il pas celui qui affirmait vouloir « une société de confiance », en précisant que, pour cela, une seule loi ne saurait suffire ? collègues, malgré cette déception, la commission spéciale et le Sénat dans son ensemble ont fait preuve de leur capacité à rebondir, pour créer les conditions d'un travail législatif fructueux en enrichissant, en précisant et, là où c'était nécessaire, en élaguant le Nous nous sommes réapproprié ce texte sur la confiance et nous avons fourni un travail considérable. Bien sûr ! À ce titre, permettez-moi d'abord de remercier tout particulièrement les rapporteurs, Pascale Gruny et Jean-Claude Luche, et tous les membres de la commission spéciale de leur contribution. En perfectionnant les dispositifs, en améliorant des rédactions souvent complexes et en retirant certains des éléments les moins pertinents, nous avons contribué à produire un texte de loi meilleur. Je citerai, à cet égard, quatre apports importants du Sénat du Sénat : la reconnaissance, au bénéfice des collectivités locales, dans leurs relations avec l'État, d'un droit à l'erreur ; la possibilité d'une validation expresse des points examinés lors d'un contrôle fiscal ; la limitation de la durée cumulée des contrôles administratifs sur les très petites entreprises à six mois sur une période de trois ans enfin le maintien du recours à l'enquête publique plutôt qu'une simple procédure de consultation par voie électronique préalablement à l'autorisation d'un certain nombre de projets agricoles. L'examen de ce texte a également été l'occasion de recourir pour la première fois à la procédure de législation en commission. Celle-ci nous aura permis d'accélérer significativement nos travaux en séance publique sans que le débat perde en qualité. Plusieurs d'entre vous, initialement sceptiques quant au recours à cette procédure, l'ont saluée à l'issue de nos travaux. Avec cette nouvelle procédure, le Sénat est pionnier, et c'est tant mieux : pour ceux qui pensent que le bicamérisme serait d'un autre temps ou que le Sénat est la maison des conservatismes, il faudra repasser ! Très bien Avec cette innovation, nous affirmons la capacité du Sénat à s'adapter, à légiférer sur des sujets plus techniques, avec un vrai travail de fond en commission, un travail de qualité bien sûr. Ce travail obéit néanmoins à un préalable le pacte de confiance et d'intelligence partagées, contrepartie du droit de veto. Mes chers collègues, je vous invite à voter ce projet de loi qui, malgré ses défauts, contribuera à moderniser les rapports des Français avec leurs administrations, qui doit permettre de rendre ces dernières plus performantes et plus efficaces.

Pourquoi cette position d'abstention sur un texte qui, pour faire écho à la discussion générale, vise à faciliter la vie de nos concitoyens, de nos entreprises et de nos administrations ? Nous avons posé un certain nombre de balises avec les dispositifs principaux du texte- le droit à l'erreur, le droit au contrôle, la médiation, la transaction -, mais il est vrai que c'est une impression un peu plus complexe qui domine à ce stade de la procédure. J'ai suivi l'intégralité des débats, et force est de constater que ce qui en ressort peut parfois donner le tournis. Nous avons débattu longuement et précisément d'un certain nombre de sujets, si bien que le débat n'a pas du tout été occulté.

Il est toujours curieux d'assister à l'embolie progressive de certains textes, d'un texte dont la raison d'être est de promouvoir et de permettre une plus grande simplicité, une plus grande sérénité des relations administratives. La fameuse formule de Michel Crozier « on ne change pas la société par décret » s'applique aussi au législateur. Dit autrement, l'excès de règles est parfois autant à craindre que l'absence de règles. Il est inutile d'empiler la norme sur la norme. C'est d'ailleurs l'un des grands mérites de ce projet de loi que de reconnaître que d'autres outils juridiques sont disponibles pour faire face à telle ou telle situation entre les administrés et l'administration. Ce texte s'articule avec la transformation de l'action publique. C'est en effet demain aux agents publics qu'il reviendra de l'appliquer. Il reviendra notamment aux managers et aux gestionnaires des ressources humaines de permettre au droit à l'erreur de pleinement se déployer. Car derrière la législation, il y a des agents publics qui ne demandent qu'à pouvoir accomplir sereinement un service public de qualité. Ce sont les agents publics qui feront vivre au quotidien cette administration qui conseille, cette administration qui dialogue

Longtemps la confiance a été la grande absente des relations entre l'État et celles et ceux qui le font fonctionner. Ce texte pose un jalon, il envoie un signal. Il montre aux agents publics du terrain que leurs retours, leurs initiatives, leurs difficultés sont des leviers d'amélioration du service public.

Ce texte est un appel à une société plus confiante, plus sereine, qui offre de nouvelles respirations aux relations entre les administrations et l'usager. Puisse cette sérénité inspirer les travaux de la commission mixte paritaire.

citoyen et écologiste. Selon la légende, avant la visite de Catherine II en Crimée, le Premier ministre d'alors, Grigori Potemkine, aurait donné l'ordre de cacher la misère des villages traversés par l'impératrice derrière des façades de carton-pâte. Il n'était pas Premier côté façade, on institue rien de moins qu'une société de confiance en mettant l'État à son service ; côté arrière-cour, on entasse un bric-à-brac de dispositions disparates, sans lien entre elles, voire sans lien avec l'objectif. présent, les sommets de l'État avaient pensé soigner la sécession civique des Français par la transparence. On expérimente donc une nouvelle médecine : la confiance. Rien ne sera possible sans cette relation de confiance et de responsabilité » déclinait il y a déjà quelques mois Emmanuel Macron dans son discours-fleuve du congrès de l'Association La transparence s'était faite sur le dos des élus ; la société de confiance sera réalisée sur celui de l'administration. Curieux mélange de théorie du, du soin, chère aux sociaux libéraux du et de et de populisme chic : calmer la défiance des citoyens en transformant une administration jugée soupçonneuse, tatillonne, voire hostile en administration de l'accueil. L'administration publique n'administre plus, elle donne des conseils et rend des services. Son objectif est non plus de concilier l'efficacité et l'équité de traitement des citoyens, mais de leur donner confiance dans leur administration, donc en eux-mêmes. C'est d'abord un service social. C'est une administration qui accompagne, qui reconnaît le droit à l'erreur et qui prévient celle-ci, le tout, bien sûr, avec des moyens en voie de réduction. Côté contenu, on est loin du compte. Le produit phare, le droit à l'erreur pour les personnes de bonne foi ayant méconnu pour la première fois une règle, se borne largement à inscrire dans la loi des pratiques existantes qu'un décret, voire quelques circulaires, aurait suffi à généraliser. revanche, ce texte laisse intacts les dilemmes de la vie réelle : la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration qui doit démontrer une volonté de méconnaître délibérément la règle. Mais comment démontrer une intention ? Être contrôlé devient un droit, mais un droit que l'administration peut refuser s'il a pour effet de « compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité de mener à bien son programme de contrôle. Quant à la limitation expérimentale des contrôles des petites et moyennes entreprises, les PME, elle ne concerne ni les contrôles relatifs au respect des règles européennes, à la préservation de la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à l'environnement ni les contrôles résultant de l'exécution d'un contrat ou effectués par une autorité de régulation. Elle n'est pas non plus opposable quand existent « des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire. » On

Même perplexité quant au certificat d'information et au référent unique. Le certificat d'information engage la responsabilité de l'administration : clair et précis, il sera la source de multiples plaintes et contentieux ; se limitant à des généralités, il sera inutile. Quant au référent unique, où trouvera-t-on ces encyclopédies vivantes ? Mystère ! L'autre moitié du texte se partage entre la reprise de vieilles lunes et celle des habituelles propositions de loi portant diverses dispositions de modernisation et de simplification de ceci ou de cela.

Autre vieille lune, la stimulation de la construction par l'innovation, sans trop se soucier des conséquences en termes de sécurité publique, de sécurité tout court et de protection de l'environnement. puis on voit ! C'est ce qu'on appelle remplacer une logique de moyens par une logique d'objectifs. Pour les résultats et les contentieux, comme pour la revalorisation des retraites agricoles, il faudra attendre. Pour le reste, au détour des articles, on ne révise rien de moins que la loi de 1905 sur la séparation des Églises et l'État, le code minier, le code de l'action sociale et des familles, le code de la consommation, le code monétaire et financier pour protéger les banques des recours de leurs emprunteurs, le code de l'éducation et la réglementation des cirques- j'ai dû en oublier. Que penser d'un tel projet de loi, sinon que l'on se moque du Parlement ? La mission de ce dernier n'est ni de participer aux campagnes promotionnelles de l'exécutif, ni de se dessaisir, sauf exception, de son pouvoir de légiférer au profit de celui-ci, ni, inversement, de diriger l'administration. Sa mission est de faire des lois qu'on n'aura pas à réviser dès que votées- à l'inverse de celle-ci.

avant d'évoquer le texte en lui-même, permettez-moi de revenir sur la procédure qui a permis son élaboration- je veux parler de la législation en commission. Procédure nouvelle, innovante, et finalement concluante, cette méthode, sur les sujets techniques qui nous intéressaient, a fait ses preuves. Offrant un gain de temps indéniable en séance publique, elle aura permis d'approfondir le débat sur d'autres points qui, sans être dépourvus de toute technicité, présentaient une plus grande acuité. Hasard du calendrier, le texte pour lequel cette procédure fut inaugurée porte sur la confiance. Or cette procédure est un pacte de confiance du Parlement envers ses membres et de ses membres envers leurs commissions. Après ce premier succès, elle a vocation à prospérer. Il s'agit là d'un utile renouveau de la procédure législative, et force est de constater que c'est du Sénat que cette innovation émane. Nous pouvons en être fiers. projet de loi aussi complet que complexe, et avec l'utilisation donc d'une procédure nouvelle, nous devons saluer la sagacité de la commission spéciale, de son président

Certaines dispositions demeuraient en effet imprécises, et conséquemment délicates à mettre en oeuvre. Ce n'est plus le cas. Les douze articles examinés la procédure de législation en commission, ainsi que les nombreux articles seulement modifiés par les amendements de la commission spéciale ont été substantiellement améliorés. Cet important travail de la commission spéciale, sur le plan tant quantitatif que qualitatif, est à souligner. Le travail en commission fut important, le travail en séance publique le fut tout autant, et le texte- à présent renommé « projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public » -comporte treize nouveaux articles,

La taille du texte se justifie en effet par son objet même et par la transversalité qu'il implique. L'administration est au coeur du fonctionnement de notre société ; en renforcer l'efficacité impliquait nécessairement une multiplicité de sujets de débat. Je veux à présent évoquer le fond du projet de loi. Tout d'abord, le droit à l'erreur, qui est l'un des fondements de ce texte. Son champ d'application a été étendu aux collectivités territoriales par la commission spéciale sénatoriale. En tant que représentants des collectivités territoriales, nous devons nous réjouir de cette extension. Comme j'ai déjà pu le dire, la confiance réciproque entre l'État et les collectivités territoriales est plus que nécessaire. Avec l'extension du droit à l'erreur, cette mesure revêt une importance plus grande encore. Mais ce droit à l'erreur a également été étendu, en séance publique, à certaines règles issues du droit européen, notamment la politique agricole Ainsi, nos agriculteurs, qui travaillent dur, mais se retrouvent parfois englués dans des démarches administratives complexes, n'auront plus à craindre d'être sanctionnés alors qu'ils étaient de bonne foi. Quant à l'environnement, cette extension procède du bon sens en cette période de prise de conscience générale. Je profite également du temps qui m'est accordé pour saluer Hervé Maurey, grâce à qui a été accrue la traçabilité des flux financiers pour ce qui concerne la construction des lieux de cultes. La mesure adoptée par le Sénat permet en effet de soumettre à l'élaboration d'un plan de financement prévisionnel certifié par un commissaire aux comptes tout projet de construction d'un édifice du culte. La confiance devant en ce domaine passer par le contrôle et la transparence, nous nous félicitons de l'adoption de l'amendement à l'origine de cette disposition. Enfin, je reviendrai brièvement sur la renégociation des tarifs de rachat de l'électricité produite en mer souhaitée par le Gouvernement. Ce sujet a provoqué de vifs débats au sein de la Haute Assemblée, chaque option présentant ses avantages et ses inconvénients. Au sein même de mon groupe, des désaccords existaient, mais parce que rien ne sert plus la démocratie que le débat d'idées, je me réjouis de l'existence de ces discussions. Conformément à l'avis de la commission spéciale, la sagesse du Sénat a tranché

de loi fait preuve de bon sens ; nous nous rangerons donc à la majorité en le votant. Les idées qu'il véhicule sont les bonnes. Toutefois, nous ne nous reposerons pas sur cet acquis, car si l'ambition est grande, nous ne sommes pas encore à son niveau. Ce jalon, aussi nécessaire soit-il, n'est jamais que la première étape vers la restauration du lien de confiance qui doit exister entre l'administration et ses interlocuteurs. Aussi veillerons-nous à ce que les décrets d'application soient bien pris et à ce que les expérimentations fassent l'objet des évaluations prévues, afin que notre engagement ne soit pas vain. L'amélioration générale de notre administration doit être effective. Ce sera le sens de notre vote. La parole

Je me félicite d'ailleurs que le Sénat donne à ce texte un nom plus conforme à la modestie qui est la sienne en l'intitulant projet de loi « renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public ». de loi, le groupe socialiste et républicain l'a abordé avec enthousiasme. C'était pour nous l'occasion d'aller plus loin dans le travail de simplification législative et de modernisation de l'État amorcé par MM. Warsmann et Mandon, pour ne citer qu'eux. Mais c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme vous le savez. À l'heure du bilan, je constate que des mesures intéressantes nous sont effectivement soumises aujourd'hui. Je pense bien évidemment à l'article 2, qui instaure un droit à l'erreur qui devra permettre à nos concitoyens, sous réserve qu'ils soient de bonne foi, d'éviter des sanctions de l'administration au premier manquement.

afin que nos concitoyens éloignés du numérique ne soient pas pénalisés. Le Sénat a apporté de nombreuses contributions à ce texte, ce qui constitue une belle illustration des vertus du bicamérisme. Ma collègue Michelle Meunier et la rapporteur ont ainsi dénoncé l'habilitation à prendre par ordonnance toute mesure facilitant l'implantation, le développement et le maintien de modes d'accueil de la petite enfance. La vie quotidienne de près de 900 000 enfants accueillis, de leurs parents et des professionnels qui travaillent dans ces structures mérite mieux que le recours aux ordonnances, et la commission spéciale a eu raison de supprimer l'article 26 . Mon groupe se félicite également du renforcement des modalités de consultation du public lors de la création d'installations classées pour la protection de l'environnement. La navette parlementaire n'a cependant pas réussi à gommer certains aspects plus gênants de ce texte qui tiennent pour beaucoup à sa conception. Comme d'autres avant moi, je qualifierai ce projet de loi de fourre-tout. Ce texte comporte de trop nombreuses habilitations, procédure dont le Gouvernement abuse par un goût excessif pour le contournement du Parlement. Concernant le numérique, l'article relatif à la dématérialisation permet aux administrés de faire des démarches depuis leur domicile, ce qui leur fera gagner beaucoup de temps. Cependant, en refusant notre amendement qui visait à un accompagnement numérique des personnes les plus vulnérables, vous niez, monsieur le secrétaire d'État, la fracture numérique qui peut exister. En ne reversant pas les économies réalisées par la dématérialisation au profit d'un accompagnement des plus vulnérables, vous passez à côté d'une amélioration qui aurait rassemblé ailleurs, comment passer sous silence l'incontournable question des moyens ? Ce texte, ce n'est pas le conseil à la place du contrôle, c'est le conseil et le contrôle. L'un ne remplace pas l'autre. C'est donc davantage de travail pour les services de l'État, dans un contexte de réduction drastique des effectifs de fonctionnaires. Bien qu'il y soit peu fait mention des agents de l'État,

Enfin, le groupe socialiste et républicain signifie son opposition à l'exclusion des associations cultuelles des registres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique. Cette décision n'a aucun sens quand on se rappelle le poids des cultes lors du débat sur le mariage pour tous ou quand on observe la préparation des débats sur la bioéthique. Nous respectons les religions, mais nous attendons qu'elles participent au débat public dans la plus grande transparence.

sous réserve, et c'était le cas, d'un travail précis de définition de son périmètre. Cette PLEC démontre la capacité d'adaptation du Sénat, qui n'attend pas le Gouvernement pour réinventer le travail parlementaire. Partis enthousiastes, Partis enthousiastes, mais rapidement devenus timorés, les sénateurs socialistes s'abstiendront donc lors du vote final sur ce projet de loi.

auxquelles le Gouvernement est particulièrement attaché, soit qu'il les ait introduites dans le projet de loi présenté au Parlement, soit qu'il en ait soutenu l'adoption à l'Assemblée nationale ou dans cette enceinte, ont pu être revues, parfois même supprimées ; d'autres ont

accusant de tous les maux les valeurs fondamentales de notre République : la liberté, l'égalité, la fraternité, sans oublier la laïcité. Mon groupe tient à faire une mise au point après la publication, aujourd'hui, de l'appel de 100 personnalités contre la volonté séparatiste de certains mouvements islamistes. La liberté d'expression subit des attaques incessantes et croissantes, en particulier sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, des associations laïques sont la cible d'activistes sur des médias comme Wikipédia, Twitter ou Facebook. La gouvernance de ces supports est dépassée par ces attaques d'un nouveau genre face auxquelles nous sommes démunis. Ne nous y trompons pas, ce sont des tentatives pour déstabiliser notre modèle républicain et diviser nos concitoyens en jouant sur les difficultés qu'ils traversent au quotidien. C'est pourquoi le groupe du RDSE veut rappeler combien il est attaché aux valeurs de notre République. Oui, la liberté est la même pour chacun dans notre pays. Oui, l'égalité entre tous, femmes ou hommes, est la loi. Oui, la fraternité est un pilier de notre République, faite d'humanisme et d'universalisme. Oui, la laïcité est le ciment de ces principes républicains, tout comme la loi de 1905, qui instaure la neutralité de l'État et sépare son organisation de celle des cultes. Bien que les intégristes de tous bords tentent de discréditer la laïcité, nous rappelons qu'elle ne stigmatise aucune religion, aucun croyant, aucun non-croyant, et qu'elle garantit l'égalité de traitement de tous nos concitoyens.

Je pense que nous devons la défendre, l'expliquer. Nous devons expliquer à ceux qui doutent encore de son sens ou souhaitent le remettre en cause, et à ceux qui font mine de l'ignorer qu'elle est un principe de liberté-

présenté, à l'occasion d'un comité interministériel qui se déroulait à Lille, un ensemble de mesures pour prévenir la radicalisation

et engagée vers le progrès social, une mesure qui va enfin mettre un terme à la précarité de l'emploi et à la situation terrible de celles et ceux qui en sont privés. J'ai en effet appris ce matin que vous alliez renforcer les contrôles et les sanctions à l'égard des chômeurs. à l'égard des chômeurs. Quelle audace ! Il faut en avoir du courage politique pour s'attaquer ainsi aux catégories les plus fragiles de la population. Les cas de fraude qui requièrent, selon vous, que l'on triple les effectifs chargés du contrôle concernent près de 5 % des prestations versées et 0,4 % des demandeurs d'emploi. Un véritable fléau, assurément ! Surtout en comparaison des 60 à 80 milliards d'euros de fraude fiscale, sans compter toutes les techniques d'optimisation que les grandes entreprises et autres fortunes de ce pays mettent en oeuvre grâce à leurs avocats spécialisés. Avec vous, madame la ministre, toute personne n'acceptant pas n'importe quel travail, même précaire, sous-payé, situé à une heure de chez elle, devra être radiée, alors que les employeurs ont, quant à eux, un droit à l'erreur, une fiscalité avantageuse et un pouvoir renforcé dans l'entreprise. Pour appuyer votre mesure, le patronat nous dit que certains secteurs manquent de main-d'oeuvre, mais sans jamais remettre en question les conditions de travail et les salaires proposés. Évidemment, pas de mépris de classe, pas de culpabilisation des « privés d'emploi » ..., mais ce simple qualificatif est déjà en lui-même stigmatisant ! Or, rappelons-le, une personne

Monsieur le Premier ministre, alors que l'économie française crée de plus en plus de richesses, ce dont chacun peut se réjouir, les Français ne peuvent ni entendre ni comprendre votre refus de mieux les répartir. Quelles

le Parlement. Plus de 12 millions de Français, c'est-à-dire un Français sur cinq, souffrent de précarité énergétique. Jeunes et étudiants, retraités ou familles monoparentales, ils vivent dans de véritables passoires thermiques et consacrent 10 % de leurs revenus aux dépenses énergétiques. Face à cette situation alarmante, les gouvernements successifs se sont mobilisés. Depuis le 1 janvier, un chèque énergie est proposé aux ménages dans le besoin pour les aider à payer leurs factures, remplaçant ainsi les tarifs sociaux de l'énergie. Le montant de ce chèque s'élève en moyenne à 150 euros par an. Or certains locataires payent jusqu'à 320 euros par mois pour maintenir la température de leur logement à 18 degrés. Le plan quinquennal de rénovation thermique de 500 000 logements par an à compter de 2017 vise à améliorer la situation économique et sanitaire de ces foyers. Mais quand bien même ces engagements seraient tenus, ils s'appuient, pour le parc privé, sur des mécanismes volontaristes de crédits d'impôt, de prêts et de certificats d'économies d'énergie. Une question reste ouverte : les citoyens les plus vulnérables, les jeunes, les retraités, les familles monoparentales mobiliseront-ils volontairement ces aides ? Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur la responsabilité sociétale des acteurs privés du secteur de l'énergie dans la détection et l'accompagnement des foyers énergétiquement précaires. En effet, les opérateurs privés de distribution d'énergie ont effectué plus de 300 000 interruptions ou résiliations de fourniture d'électricité ou de gaz en 2016. Ces mêmes opérateurs déploient des compteurs communicants dits intelligents sur l'ensemble du territoire et sont détenteurs d'une manne de données de consommation qu'ils pourraient valoriser dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. Qu'en est-il de l'implication de ces entreprises assurant une mission de service public dans la prévention, la détection et l'accompagnement de ces foyers en difficulté ? La parole

L'expérience avait été tentée dans quatre départements. Nous avons décidé qu'elle serait généralisée à l'ensemble du territoire. Le deuxième niveau d'action, vous l'avez dit,

La ville kurde d'Afrin, au nord de la Syrie, est tombée dimanche aux mains des forces turques et de leurs alliés. Afrin était encerclée depuis mardi, 250 habitants ont fui et, une fois de plus, c'est à une véritable catastrophe humanitaire que nous avons assisté. Le résultat,, de cette opération militaire turque est double : d'une part, la zone a fait l'objet du nettoyage ethnique que l'on craignait ; d'autre part, le combat mené par les Kurdes contre Daech s'en trouvera, bien entendu, ralenti. Pis, le président Erdogan a annoncé hier qu'il ne comptait pas en rester là. Son objectif assumé et affiché est de reconquérir la région frontalière pour y remplacer les populations kurdes. La France, jusqu'à présent, soutenait les Kurdes syriens dans leur combat contre Daech. Le président Hollande, en son temps, avait décidé d'intervenir à Kobané, entraînant avec lui les Américains et les forces de la coalition. La France était alors sans ambiguïté aux côtés des Kurdes, combattants bien seuls, au départ, contre le terrorisme islamique ; on l'a oublié. La discrétion du président Macron, tout au long de cette peu banale opération militaire turque, correspond-elle à un renversement de stratégie Les Kurdes seraient-ils soudain devenus aux yeux de la France des terroristes, alors qu'ils étaient hier nos alliés ? Et quel message la France envoie-t-elle au monde en se révélant incapable de venir en aide à ses alliés, alors même que ceux-ci ont besoin de nous ?

la chute d'Afrin dimanche, après deux mois d'offensive turque, marque une nouvelle escalade dans la tragédie que connaît la Syrie. Vous l'avez dit, c'est un nouveau coup porté à une situation humanitaire déjà catastrophique des dizaines de milliers de personnes sont déplacées ; celles qui restent se trouvent dans une situation critique, privées d'eau, d'électricité et de secours. C'est aussi un coup porté- vous l'avez dit, monsieur le sénateur -à la campagne contre Daech, à laquelle les forces démocratiques syriennes ont apporté une contribution décisive. La France en a pleinement conscience, la France ne l'oublie pas. Cela ne suffit pas, Daech n'est toujours pas vaincu en Syrie. C'est enfin un coup porté à la trêve humanitaire décidée par la résolution 2401 du Conseil de sécurité des Nations unies qui exige une cessation des hostilités sur l'ensemble du territoire syrien. La position de la France est constante. Les préoccupations de la Turquie concernant la sécurité de sa frontière ne doivent pas la conduire à une implantation militaire dans la profondeur du territoire syrien. Nous ne ménageons pas nos efforts pour une désescalade des tensions dans le nord de la Syrie. La preuve ! Dans l'immédiat, la Turquie doit aussi assumer ses responsabilités, faire cesser les pillages et les violences, ... Et l'implantation des groupes radicaux et assurer le libre retour dans des conditions de sécurité de la population civile déplacée. Blabla ... Il faut aussi qu'une gouvernance représentative de l'ensemble des composantes de la société locale et de leurs aspirations soit mise en place. Je le répète, seule une solution politique inclusive, c'est-à-dire incluant aussi les Kurdes, ... Quelle honte ! ... est à même d'assurer la stabilité de la Syrie et la sécurité de ses voisins, dont la Turquie.

Il le sait, la Ford Motor Company a annoncé le 27 février dernier qu'elle renonçait à confier à Ford Aquitaine Industries la fabrication d'une nouvelle transmission automatique à huit vitesses, ce qui aurait donné du travail aux salariés pendant plusieurs années. Ce bassin d'activité, vital pour la Gironde et la métropole bordelaise, est donc menacé de fermeture dès 2019. Cette fermeture concerne près de 1 000 emplois directs et 4 000 emplois indirects. Le groupe Ford a perçu des millions d'euros d'aides publiques, notamment 14 millions lors de la signature de la dernière convention. M. le ministre de l'économie et des finances avait alors immédiatement réagi à cette désastreuse annonce et qu'il avait reçu différents responsables politiques, ainsi que les représentants des syndicats. À la suite de ces rencontres,

Monsieur le sénateur Alain Cazabonne, je répondrai à la place de Bruno Le Maire, qui participe actuellement au G20 en Argentine, mais s'est bien sûr personnellement occupé du sujet que vous évoquez. Ce sujet est douloureux. En effet, le groupe Ford a annoncé le 27 février dernier sa décision de ne pas investir pour assurer l'avenir du site de Blanquefort, qui compte près de 1 000 salariés. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle, que nous déplorons. Bruno Le Maire a eu l'occasion de le dire au président de Ford Europe, il a tenu une réunion de crise avec les représentants des salariés et les élus concernés dès le 2 mars dernier. Il a obtenu que Ford maintienne le niveau des charges de l'usine jusqu'à la fin de 2019. Il faut mettre à profit ce délai pour chercher des solutions durables pour le site. Pour l'État comme pour les salariés, le premier responsable de la pérennité du site de Blanquefort est le groupe Ford lui-même, qui, à ce jour, est bénéficiaire. C'est à Ford de proposer des solutions permettant d'assurer la pérennité de ce site industriel et de garantir que d'éventuelles restructurations qu'il pourrait décider soient menées de manière parfaitement responsable. Il ne faut pas réitérer la mauvaise expérience de 2011, lorsque Ford avait tenté de céder le site à un industriel trop peu solide, puis avait été obligé de le reprendre quelques mois plus tard. Un groupe de travail de haut niveau a été constitué avec la direction de Ford et le délégué interministériel aux restructurations, M. Jean-Pierre Floris. Des comités trimestriels vont se tenir avec les salariés et les élus, à l'invitation du préfet. Le 5 avril prochain, M. Floris se rendra chez Ford Europe, afin de discuter de façon très détaillée des mesures qui seront prises pour assurer la tenue de l'engagement de charges jusqu'à la fin de 2019, et ce dans les détails les plus techniques et opérationnels.

Comme ce travailleur, des milliers de frontaliers de mon département ont été, contre leur gré, rattachés au système français d'assurance maladie et connaissent depuis des situations de double affiliation. Alors qu'ils sont contraints de cotiser deux fois, beaucoup ne bénéficient d'aucune couverture maladie et se voient, dans le même temps, réclamer des sommes importantes par les services des URSSAF. URSSAF. L'arrêt de la Cour de cassation suscite l'espoir de ces travailleurs puisqu'il dispose qu'un frontalier affilié en Suisse ne peut être affilié au régime français et doit en être radié s'il en fait la demande, peu importe l'antériorité de son affiliation au régime français. Cet arrêt règle potentiellement les milliers de situations similaires encore pendantes aussi ma question est simple. Madame la ministre, alors que vous avez hérité de cette situation complexe, vous avez l'occasion aujourd'hui de donner l'exemple de la société de confiance dont nous débattions encore la semaine dernière dans notre assemblée en adoptant le droit à l'erreur. Pour ce faire, entendez-vous tirer, dès aujourd'hui, toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation, en demandant l'abandon immédiat des procédures en cours à l'encontre des travailleurs frontaliers concernés, leur radiation de l'assurance maladie française et le remboursement des cotisations versées indûment au titre de celle-ci

concernant la situation de double affiliation de certains frontaliers travaillant en Suisse. La Cour a rejeté le pourvoi formé par la CPAM de Haute-Savoie, considérant notamment « que que la personne résidant en France qui est affiliée à l'assurance maladie obligatoire en Suisse au titre de l'activité qu'elle exerce dans cet État, ne peut être affiliée au régime français de sécurité sociale ou, en tout cas, doit en être radiée dès qu'elle le demande, peu important l'antériorité de son affiliation au régime français L'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 ne prévoyait pas de dispositions relatives à la rétroactivité. Ainsi, une majorité des frontaliers qui se sont affiliés antérieurement à cette date ont saisi les tribunaux des affaires sociales, souhaitant voir leur radiation effective à la date de leur affiliation en Suisse. La Cour de cassation a tranché ces contentieux en leur faveur. À ce jour, 9 789 recours sont en instance auprès des tribunaux des affaires de de sécurité sociale, les TASS, dont 9 708 au TASS de Mulhouse et 75 devant les cours d'appel. Afin de solder cette situation et souhaitant rassurer l'ensemble des frontaliers, les autorités compétentes françaises vont demander à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de prendre en compte la décision de la Cour de cassation en reconnaissant la radiation à la date d'affiliation en Suisse, en restituant les cotisations sociales perçues sur la période considérée ... Très bien ! ... et en abandonnant les mises en demeure auprès des frontaliers qui ne s'étaient pas acquittés de leurs cotisations. Comme vous le constatez, madame la sénatrice, l'État s'engage et l'État assume ! Très bonne

Depuis quelques années, la mission de l'aide sociale à l'enfance assurée par les conseils départementaux évolue. Une part croissante des situations concerne les mineurs non accompagnés. En Loire-Atlantique, leur nombre est passé de 50 en 2012 à près de 500 en 2017 ; il a décuplé en cinq ans, doublé en un an, comme au plan national.

Lorsque la minorité et l'isolement sont reconnus, les jeunes issus de parcours migratoires pénibles, faits d'épreuves, d'errances et de souffrances, sont accueillis en vertu de la protection que nous leur devons. À l'automne, votre gouvernement semblait avoir entendu les demandes de soutien exprimées par l'Assemblée des départements de France, l'ADF. Le budget pour 2018 accordait un financement exceptionnel. En janvier dernier, le Conseil national de la protection de l'enfance invitait l'État à prendre la responsabilité de la mise à l'abri et de l'évaluation, au titre de ses politiques régaliennes et pour permettre aux départements d'assurer correctement la protection de ces mineurs, au nom du droit commun. Lundi dernier, votre négociation avec l'ADF a écarté cette idée de reprise, ce qui est très regrettable. Pis, elle n'a pas abouti sur la question financière. Les collectivités locales assurent ne plus pouvoir affronter seules cette situation.

Le Premier ministre a annoncé à l'automne dernier que l'État s'impliquerait davantage dans le financement de l'évaluation et de l'hébergement d'urgence des personnes se déclarant mineures jusqu'à ce que leur minorité soit confirmée. Nous travaillons à rendre plus efficace la phase d'évaluation de la minorité, notamment les vérifications qui relèvent clairement de la responsabilité de l'État. J'ai assisté moi-même à une réunion chez le Premier ministre, avec les représentants de l'Assemblée des départements de France la semaine dernière. Le dialogue est en cours. Nous avons fait des propositions aussi bien techniques que financières. Vous avez rappelé de l'enveloppe d'urgence. Je crois qu'il faut aussi essayer de trouver, et c'est l'objectif du Premier ministre, un accord qui soit pérenne. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour le groupe Les Républicains.

à la suite de l'arrêt des négociations sur la convention nationale des chirurgiens-dentistes, une procédure d'arbitrage avait été mise en oeuvre en 2017. Ce règlement arbitral cristallisait les tensions des différents syndicats libéraux. Aussi, j'ai souhaité le suspendre lorsque je suis arrivée au ministère. Notre impératif est avant tout de répondre aux besoins légitimes des Français en matière de santé, de prévention et d'accès aux soins. En matière de santé et de prévention, les maladies bucco-dentaires peuvent favoriser l'apparition, la progression ou l'aggravation de certaines maladies générales. Il est donc important que les chirurgiens-dentistes s'intègrent mieux dans les parcours de soins et de santé, en lien avec les autres professionnels de santé, et que les soins conservateurs soient revalorisés. En matière d'accès aux soins, nous nous devons de mettre en oeuvre la promesse du Président de la République : le reste à charge zéro concernant les prothèses dentaires. Des négociations sont donc en cours avec la profession des chirurgiens-dentistes dans le cadre de la négociation conventionnelle. Cela ne pourra pas se faire sans un dialogue constructif prend un certain temps, mais il avance. En concertation avec les trois syndicats représentatifs, ces négociations conventionnelles ont été rouvertes cette année avec trois objectifs principaux : l'accès financier aux soins, le développement de la prévention et une attention particulière aux besoins des publics les plus fragiles. Il est primordial de responsabiliser l'ensemble des acteurs, afin de parvenir à diminuer le reste à charge sur les prothèses dentaires, tout en valorisant le travail de prévention primaire et secondaire des chirurgiens-dentistes. Les évolutions à venir modifieront durablement- nous le souhaitons -la pratique des soins dentaires en France, dans l'intérêt des patients et des professionnels. La parole

comme c'est le cas en Espagne, et que le reste à charge soit une usine à gaz dont l'administration a parfois le secret. Nous souhaitons que les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers et quelle que soit leur spécialité, soient vraiment entendus et que vous les écoutiez, car ce sont eux qui exercent cette profession. Il y va aussi d'un maillage territorial équilibré sur le territoire !

Ma question s'adresse à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur. Le Président de la République a récemment annoncé qu'il comptait reprendre le dossier de l'organisation de l'islam en France. Le 14 mai prochain débuteront les célébrations du ramadan. À cette occasion plusieurs centaines d'imams, psalmodieurs, récitatrices arriveront du monde entier en France, certains avec des conventions, d'autres uniquement avec des visas de tourisme.

et le financement de l'islam dans notre pays. Effectivement, la France accueille tous les ans des imams qui sont souvent formés dans les pays du Maghreb.

Ce dispositif permet de s'assurer que les imams ont un certain niveau de formation et qu'ils parlent français. Cela dit, comme vous l'avez indiqué, le Président de la République a lancé un chantier sur l'islam de France.

sur ces sujets depuis Bernard Cazeneuve et l'instance de dialogue. Il faut vraiment, je le crois, travailler sur ces questions pour le respect et la sécurité de tous, et notamment de nos concitoyens de confession musulmane, de façon qu'ils puissent exercer leur culte dans les meilleures conditions.

La politique de la ville, ce sont quarante années de combat et de mobilisation. La politique de la ville, ce sont des moyens spécifiques de l'État dans les quartiers dits prioritaires, pour réduire les inégalités sociales entre les territoires. Développement économique, éducation, emploi, rénovation urbaine, cadre de vie sont autant de domaines d'action engagés pour améliorer les conditions de vie de ces habitants. ans, beaucoup a été réalisé par les gouvernements qui se sont succédé : zones d'éducation prioritaire, missions locales, Agence nationale pour la rénovation urbaine, entre autres. Pourtant, le chômage dans ces quartiers reste deux fois supérieur à la moyenne nationale et le sentiment de relégation est vif. Il est plus qu'évident que la politique de la ville a encore de nombreux défis à relever. Le Gouvernement s'est donné comme objectif de réduire de 50 % l'écart de taux de chômage entre les quartiers et la moyenne nationale sur cinq ans et d'améliorer d'une manière générale le cadre de vie de ces habitants. Des mesures spécifiques ont d'ores et déjà été décidées : la création des emplois francs ; le doublement du nouveau programme national de rénovation urbaine ; le développement des conseils citoyens pour associer la population ; le dédoublement des classes de CP en REP+. Malgré l'engagement des acteurs sur le terrain et les progrès réalisés en matière de cohésion sociale et d'emploi, le regard porté sur les quartiers populaires reste encore trop souvent négatif et stéréotypé. Dans mes fonctions mayorales antérieures, j'ai pu mesurer la persistance de ces préjugés. Si ma commune a bénéficié positivement de la politique de la ville, j'ai pu aussi constater les carences des différentes politiques qui se sont succédé. s'il y a eu de formidables succès, tels que les plans de rénovation urbaine, si des territoires se sont transformés, il y a eu aussi des échecs, des coups d'arrêt. Le défi de la politique de la ville est toujours et encore immense. C'est celui de territoires qui ont concentré toutes les difficultés, avec un chômage de masse qui s'y est installé depuis parfois plusieurs décennies. Dans ce cadre, rien n'est plus important que de reconnaître et de valoriser les contributions de la société civile, et d'engager une nouvelle étape reposant sur une politique de droit commun de l'État et des collectivités.

pouvez-vous nous livrer un point d'étape sur la feuille de route du Gouvernement et rassurer ainsi les acteurs d'un dossier essentiel pour garantir la promesse républicaine ?

votre question dresse un bilan objectif et réaliste de la situation dans ces quartiers. Ce que je veux dire de manière liminaire, c'est qu'il ne faut en aucun cas opposer les différents territoires. Dans notre pays, un certain nombre de territoires ont des difficultés particulières, que ce soient les quartiers prioritaires de la politique de la ville, certains territoires ruraux ou certaines villes moyennes. Il ne s'agit pas de faire jouer la concurrence des uns contre les autres s'agissant des mesures que nous devons mettre en place pour lutter contre ce décrochage, lequel ne remonte pas à quelques mois, mais est le résultat de plusieurs décennies d'évolutions sociétales et économiques. Par rapport à cette situation,

afin de finaliser un certain nombre de propositions. De la même manière, nous avons saisi dix groupes de travail au niveau national pour faire des propositions. Aujourd'hui, nous en sommes à une phase d'étape, nous n'avons pas de décisions à prendre. Nous sommes à l'écoute. D'ici à un mois, un rapport sera soumis, et nous devrons alors prendre un certain nombre de décisions. Vous avez parlé, à juste titre, de la question de l'image. Je rencontrais hier la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, pour travailler avec elle sur la définition de nouveaux moyens destinés à revaloriser l'image de ces territoires, dans lesquels il y a aussi beaucoup de belles choses. Nous avons l'impérieuse nécessité de travailler ensemble pour les mettre en valeur- c'est aussi ce que fait le Gouvernement. La parole

postes, l'ARCEP, et les opérateurs ont su, avec l'appui des collectivités et de leurs associations, sortir par le haut de la problématique de la couverture mobile. Vous le remarquerez, monsieur le ministre de la cohésion des territoires, Mais s'agissant de la desserte fixe, c'est le chemin inverse que le Gouvernement semble prendre petit à petit. Vous aviez pourtant annoncé, à la fin du mois de juillet dernier, que le besoin financier nécessaire à la poursuite du déploiement du FTTH, le réseau, par les réseaux d'initiative publique serait de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Il y avait matière à poursuivre le plan France Très haut débit qui est jusqu'alors une réussite unanimement reconnue. Or depuis cette annonce, je dois le dire, ces engagements budgétaires tardent à se concrétiser.

locaux, l'AMEL, sans autre alternative possible ; l'absence de soutien à la proposition de loi visant à sécuriser les déploiements FTTH, publics et privés, malgré un vote unanime du Sénat ; et la refonte annoncée de l'offre de montée en débit. Loin de la cohésion des territoires, on s'oriente vers une France à deux vitesses : celle qui aura accès au plan France Très haut débit et celle qui n'aura que le plan France PRM-MeD, Aussi, je souhaite savoir, monsieur le ministre, dans quels délais, dans quelles conditions financières et avec quelles limitations de montages juridiques et technologiques vous allez rouvrir le plan en vue d'assurer la réalisation des objectifs de déploiement auquel le Gouvernement a déclaré pleinement souscrire. La parole

Monsieur le sénateur Patrick Chaize, le Président de la République l'a rappelé dès les premiers jours de son mandat, la couverture nationale numérique est un enjeu essentiel. Elle est aujourd'hui le premier accès aux services économiques, aux services publics, aux services d'information, aux services de formation, aux services de communication et bientôt de santé. Face à cette révolution, aucun territoire ne peut être exclu.

couverture mobile, vous l'avez rappelé, il y a eu un changement de paradigme, je n'y reviens pas. Nous avions l'occasion, au moment de l'attribution de ces nouvelles licences, soit de penser simplement au budget de l'État, soit de penser à la fois au budget de l'État et à l'accélération du déploiement. Vous l'avez dit, cet accord va permettre un surinvestissement de plus de 3 milliards d'euros des opérateurs dans les prochaines années, ce qui nous permettra de tenir ces objectifs. Concernant la couverture fixe, la méthode était celle du changement de braquet, de l'accélération. Nous avons consolidé l'intégralité de l'engagement des 3,3 milliards d'euros du plan France Très haut débit. Nous avons mobilisé près de 300 millions d'euros, et nous avons conforté, sans jamais trembler, la signature de l'intégralité des réseaux d'initiative publique qui étaient en cours. À l'époque, vous aviez posé une question, vous inquiétant pour ces réseaux d'initiative publique. Ils sont maintenant tous sécurisés et en cours de déploiement. Pour les territoires ruraux,

des Français seront couverts en très haut débit d'ici à 2022, et pour beaucoup ce sera bien avant. La volonté de mobiliser intelligemment les ressources publiques autour des nouveaux dispositifs de l'AMEL va nous permettre de penser l'après-2022. C'est tout le dialogue qui a lieu aujourd'hui. Ce n'est pas une fermeture, c'est un engagement à penser le futur ensemble

le Président de la République a choisi la Journée internationale de la francophonie pour dévoiler son plan en faveur de la langue française. Il était urgent de passer du discours aux actes. Comment peut-on en effet se faire le chantre de la francophonie tout en coupant de 33 millions d'euros les budgets consacrés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en supprimant des postes de professeurs ? N'est-il pas contradictoire de vanter le français comme langue d'avenir et de parler anglais dans les grandes enceintes internationales, où l'on trouve pourtant d'excellents interprètes ? Alors qu'un grand plan est en train d'être dévoilé, je veux mettre en garde contre une approche trop jacobine. La francophonie ne peut plus être un instrument piloté par le Quai d'Orsay par l'Élysée. Tant que nous la concevrons comme une stratégie impulsée par Paris, nous nous couperons des pays francophones. La francophonie se construirait alors sans nous, alors que la francophonie du XXI siècle se doit d'être agile, pragmatique, en perpétuelle adaptation aux attentes locales. Il ne s'agit pas de considérations théoriques. L'indépendance du réseau de nos 834 alliances françaises est aujourd'hui menacée. Un placement sous tutelle du Quai d'Orsay ou des instituts français serait une erreur stratégique et un très mauvais signal envoyé aux francophones et aux autorités des pays où sont implantées les alliances. Le français doit sortir des sphères académiques pour redevenir la langue des secteurs d'avenir, créateurs d'emplois. Pour mobiliser l'énergie des jeunes et leur offrir de nouvelles opportunités à l'international, j'avais suggéré la création- très nécessaire -d'un volontariat international d'enseignement en français. Le grand plan pour le français du Gouvernement concrétisera-t-il

ministre chargée des affaires européennes. Madame la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam, vous l'avez dit, le Président de la République est en ce moment même à l'Académie française pour présenter la nouvelle stratégie de la France pour la promotion du français et du plurilinguisme dans le monde. Je crois que ce qu'il annonce répondra à vos attentes. vos attentes. En cette Journée internationale de la francophonie, je veux vous confirmer l'engagement du Gouvernement pour faire de la promotion de la langue française l'un des grands enjeux de ce quinquennat. Le français est parlé aujourd'hui par près de 300 millions de locuteurs dans le monde ; il pourrait l'être par plus de 700 millions en 2050. Il faut en tirer toutes les conséquences. Le français est un atout majeur de la France dans la mondialisation. C'est aussi un bien commun, au-delà des frontières hexagonales. Cela doit nous conduire à décentrer notre regard sur le français, qui est autant une langue d'Afrique et d'ailleurs que de France. Il nous faut aussi prendre la pleine mesure du défi éducatif sur le continent il nous revient de conforter notre capacité de rayonnement, notamment grâce à ces magnifiques outils, que vous avez cités, que sont les lycées, les alliances et les instituts français.

qui est des lycées français, le chef de l'État a annoncé qu'il comptait doubler le nombre d'élèves dans ces établissements à travers le monde. Nous devons relever deux défis renouveler notre capacité à atteindre de nouveaux publics, d'une part ; accélérer la prise de conscience francophone en France même, d'autre part. En cette Journée internationale de la francophonie, madame la sénatrice, de rendre hommage à votre mobilisation sur ce sujet et de saluer vos idées, notamment celle de la création d'une cité de la francophonie à Villers-Cotterêts et celle d'un volontariat international d'enseignement en français, que vous venez de rappeler. Ces deux idées viennent d'être reprises par le Président de la République ; il vient d'en faire l'annonce il y a quelques instants. Nous en

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur de la commission des lois, monsieur le rapporteur de la commission des affaires européennes, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis heureuse de retrouver votre hémicycle pour présenter, au nom du Gouvernement, ce projet de loi relatif à la protection des données personnelles, dont l'objet est d'adapter au droit de l'Union européenne la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le nouveau cadre juridique européen doit, en effet, entrer en vigueur en mai prochain. Les textes communautaires visés, qui sont l'aboutissement d'une longue phase de négociations, traduisent l'ambition très forte de notre continent dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Pionnière avec la loi du 6 janvier 1978, dont nous venons de fêter les quarante ans, la France a pris une part très active dans les négociations européennes, afin de maintenir et de promouvoir son modèle de contrôle et de protection qui constitue encore aujourd'hui une référence en Europe et dans le monde. Fruit d'un compromis, le paquet européen « protection des données » a été adopté par le Parlement européen et le Conseil le 27 avril 2016. 27 avril 2016. Il se compose de deux textes : d'une part, un règlement, qui constitue le cadre général de la protection des données, et, d'autre part, une directive, qui vise les données à caractère personnel en matière pénale. Je souhaite évoquer devant vous ces deux textes, avant d'aborder la méthode retenue par le Gouvernement pour les traduire dans notre droit et, enfin, deux problèmes politiques qui me semblent importants. me semblent importants. Le règlement crée un cadre unifié et protecteur pour les données personnelles des Européens. Il est applicable à l'ensemble des entreprises et de leurs sous-traitants, quelle que soit leur implantation, dès lors que ceux-ci offrent des biens et services à des personnes résidant sur le territoire de l'Union européenne. C'est un point très important : le droit européen s'appliquera chaque fois qu'un résident européen, quelle que soit sa nationalité, sera directement visé par un traitement de données, y compris donc par internet ou par le biais d'objets connectés, et ce quelle que soit la localisation du stockage et du traitement. Le règlement crée, dès lors, une procédure de coopération intégrée entre les autorités de protection des données des États membres, dont, pour la CNIL. C'est le gage d'une application uniforme des nouvelles obligations, sous l'égide du Comité européen de la protection des données. C'est aussi l'affirmation d'une conception européenne de la protection des données personnelles qui diffère diffère de celle qui est promue aux États-Unis ou dans d'autres États, comme en Chine. L'Europe entend, en effet, concilier les valeurs du progrès et de la garantie des droits et des libertés fondamentales, en renforçant la confiance des citoyens dans l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles, tout en offrant aux opérateurs économiques un environnement attractif. Le règlement instaure donc de nouveaux droits pour les citoyens, comme le droit à la portabilité des données personnelles. Il crée également un environnement attractif pour des opérateurs économiques plus responsables, Nous inaugurons, dès lors, une nouvelle ère dans la régulation, avec un changement de paradigme assez profond : il s'agit désormais, en effet, d'alléger considérablement les formalités préalables, au bénéfice d'une démarche de responsabilité des acteurs et d'accroissement des droits des individus. Ainsi, le règlement européen remplace le système de contrôle, basé sur des déclarations et des autorisations préalables, par un système de contrôle, plus plus adapté aux évolutions technologiques, fondé sur l'appréciation par le responsable du traitement des risques que présente ce dernier. Cette nouvelle approche impose aux responsables de traitement d'intégrer les exigences de la protection des données personnelles très en amont de la conception de leur produit ou de leur service et d'offrir au consommateur, par défaut, le niveau de protection le plus élevé. La désignation d'un délégué à la protection des données sera obligatoire dans le secteur public, mais des mutualisations seront possibles. possibles. Elle sera aussi obligatoire lorsque l'activité principale d'une entreprise en matière de traitement des données sensibles le justifiera. Les responsables de traitement devront également notifier les violations de données personnelles à l'autorité de contrôle, ainsi qu'aux personnes concernées en cas de risque élevé pour leurs droits et libertés. En responsabilisant les acteurs, qui devront être accompagnés par la CNIL, le projet de loi consacre également de nouvelles modalités de régulation, à travers des outils de droit souple. En contrepartie, les pouvoirs de la CNIL sont renforcés et les sanctions encourues sont considérablement augmentées, jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial consolidé.

C'est la première fois que l'Union européenne se dote d'un cadre normatif pour réglementer le traitement de ces données dans un cadre national. La directive s'applique aux traitements mis en oeuvre par une autorité compétente à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

La directive n'est en revanche pas applicable dès lors que le traitement est mis en oeuvre pour des finalités qui ne sont pas pénales ou par une autorité qui n'est pas compétente. Elle n'est pas non plus applicable aux traitements intéressant la sûreté de l'État et la défense qui ne relèvent pas du droit de l'Union européenne. Les principales innovations de la directive consistent en la création, en matière pénale, d'un droit à l'information de la personne concernée par les données personnelles traitées et en la consécration d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement. Ces droits s'exercent par principe de manière directe par la personne concernée auprès du responsable de traitement, alors que la loi actuelle prévoit un exercice indirect de ces droits pour les traitements intéressant la sécurité publique et la police judiciaire.

recèle des enjeux politiques considérables ». Le Gouvernement ainsi que le Sénat et l'Assemblée nationale en ont, me semble-t-il, saisi toute la portée. Cependant, ce texte demeure technique, car il se situe au croisement de deux textes communautaires de portée juridique distincte,

Il faudra donc, en tout état de cause, lire cette nouvelle loi de 1978 avec le règlement européen à portée de main. On peut le regretter, au regard de la complexité que cet exercice suppose, mais il en est ainsi.

Mais le projet de loi qui vous est soumis ne constitue pas seulement un exercice de transposition de la réglementation européenne. Il offre également des choix politiques, pour lesquels vous avez fait des propositions.

Conformément à la démarche de simplification des normes souhaitée par le Président de la République et à sa volonté d'éviter la surtransposition de textes européens, le Gouvernement a fait a fait le choix d'épouser la nouvelle philosophie du règlement et de supprimer la plupart des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. Ce choix a notamment été salué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il l'a également été par votre commission des affaires européennes et par son rapporteur, M. Simon Sutour, qui souligne une exploitation « mesurée » des marges de manoeuvre. Cependant, afin de ne pas affaiblir la protection des données à caractère personnel et bien que cela ne soit pas exigé par le règlement ni par la directive, le Gouvernement a fait le choix de maintenir certaines formalités préalables pour les traitements des données les plus sensibles, par exemple pour les données biométriques, les données génétiques, ou encore pour les traitements utilisant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Les Les traitements utilisant des données de santé font aussi l'objet d'un régime protecteur et unifié. Ces dispositions s'inscrivent dans la logique du maintien d'un haut niveau national de protection en la matière, conformément des résolutions européennes qu'il a adoptées en 2012 et 2013, sans faire peser de charges supplémentaires sur les petites et moyennes entreprises. Enfin, dans le champ d'application de la directive, sont également maintenues les formalités préalables à la création de tout traitement mis en oeuvre pour le compte de l'État. Par ailleurs, un point important, qui retient naturellement votre attention, doit être précisé. Le règlement fixe à seize ans l'âge à partir duquel un mineur peut consentir à une à une offre directe de services de la société de l'information, c'est-à-dire accéder aux réseaux sociaux. Le Gouvernement avait fait le choix de ne pas utiliser la marge de manoeuvre prévue à l'article 8 du règlement qui permet aux États membres d'abaisser ce seuil jusqu'à treize ans. L'Assemblée nationale a souhaité fixer cet âge à quinze ans. Votre commission des lois a décidé de supprimer cette disposition pour revenir à l'âge de seize ans.

de saisir par une norme générale des cas éminemment singuliers, surtout lorsqu'il s'agit d'identifier ce qui constitue en réalité le seuil de maturité d'un enfant. La France avait défendu le seuil de seize ans en deçà duquel l'autorisation parentale serait nécessaire pour autoriser le traitement de données Les autres pays de l'Union ont fait des choix très divers. Comme il l'avait fait lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, le Gouvernement adoptera une position de sagesse sur cette question et s'en remettra à la décision de la représentation nationale. En tout état de cause, la mise en place d'une autorisation parentale, sans lourdeur procédurale excessive, doit surtout être l'occasion de réinstaurer un dialogue au sein de la famille sur ces questions.

: âge du consentement- je viens de l'évoquer -, encadrement de l'usage des algorithmes par l'administration, renforcement des conditions de traitement des données d'infraction avec la réintroduction d'une autorisation préalable par la CNIL, ou encore introduction d'un motif de nullité contractuelle pour les fournisseurs de terminaux électroniques en cas d'installation d'applications ne respectant pas les conditions du consentement de l'utilisateur final. Nous aurons l'occasion d'en débattre dans le cadre de l'examen des amendements que le Gouvernement a déposés. Je souhaite cependant aborder deux questions : l'une est relative aux collectivités territoriales, l'autre concerne l'habilitation demandée par le Gouvernement.

Elle a adopté plusieurs amendements à leur égard : création d'une dotation communale et intercommunale pour la protection des données personnelles, mutualisation des services, suppression de la faculté pour la CNIL de leur imposer des amendes administratives, report de deux ans de l'entrée en vigueur de l'action de groupe en réparation en matière de données personnelles, encouragement de la diffusion d'informations et édiction de normes de droit souple par la CNIL adaptées aux besoins et aux moyens des collectivités ... Le Gouvernement entend parfaitement votre préoccupation- je dirais même qu'il la porte avec vous. Toutefois, il ne me semble pas juste de considérer que le Gouvernement ferait preuve d'un « mépris abyssal », comme j'ai pu le lire, à l'égard des collectivités. Notre responsabilité est bien d'accompagner les collectivités pour leur permettre d'entrer dans cette nouvelle ère dans les meilleures conditions possible. Je crois que, en la matière, il faut répondre aux inquiétudes et non pas les exacerber. Je suis certaine que telle est notre préoccupation commune. Avant même que votre commission des lois n'examine ce texte, le Gouvernement a pris la mesure de cette nécessité. Voilà quelques jours, j'ai ainsi rappelé devant les préfets, réunis place Beauvau, la nécessité d'accompagner dans cet exercice toutes les communes, notamment les plus petites d'entre elles. De même, je me suis assurée auprès de la CNIL que cette préoccupation serait effectivement prise en considération. Je tiens aussi à rappeler que les collectivités territoriales sont actuellement soumises, en tant que responsables de traitement de données, à certaines obligations, que ce soit pour assurer la gestion administrative de leur structure- je pense, par exemple, aux fichiers de ressources humaines -, la sécurisation de leurs locaux- contrôles d'accès par badge ou vidéosurveillance - ou la gestion des différents services publics et activités dont elles ont la charge. J'y insiste, car certains pourraient avoir le sentiment que nous introduisons de nouvelles obligations, alors que la philosophie du règlement européen, et donc du projet de loi, est justement fondée sur un allégement substantiel des formalités préalables, y compris pour les collectivités territoriales.

Plusieurs collectivités territoriales, dont certaines avaient déjà désigné un correspondant Informatique et libertés, se sont d'ores et déjà engagées dans cette démarche de mutualisation. Cette possibilité sera expressément rappelée dans le décret d'application sur lequel les services de la Chancellerie travaillent actuellement. Le Gouvernement s'y est engagé auprès du Conseil national d'évaluation des normes et de son président, Alain Lambert. Je veux également souligner que la CNIL mène de nombreuses actions pour aider les collectivités territoriales à respecter leurs obligations en matière de protection des données et pour les accompagner dans leur mise en conformité avec le RGPD. Elle a, par exemple, conclu avec l'Assemblée des départements de France une convention de partenariat et souhaite faire de même avec l'Assemblée des maires de France, l'AMF. De plus, la CNIL va remettre à jour le guide très complet à destination des collectivités. Je suis également parfaitement consciente des appréhensions pouvant exister quant à l'échéance du 25 mai prochain. La CNIL a donné des assurances en ce domaine et saura se montrer pragmatique, comme elle l'a été jusqu'à présent, avec les collectivités. Le Gouvernement encourage cette démarche compréhensive à l'égard des collectivités tout en insistant sur la nécessité de maintenir un haut niveau de protection des données personnelles. messieurs les sénateurs, le Gouvernement ne propose pas de revenir sur certaines avancées adoptées par votre commission des lois. Je pense, en particulier, à l'exonération des sanctions à l'égal de l'État. Le débat parlementaire- et c'est très heureux -a vocation à mettre en lumière les enjeux. De ce point de vue, le Sénat a marqué une nouvelle fois son attention aux collectivités territoriales. Il est naturel que le Gouvernement y réponde, et c'est bien tout l'intérêt de nos échanges.

Son rapporteur a estimé qu'il s'agissait de la conséquence d'une impréparation. Là encore, je crois nécessaire de rappeler quelques faits pour mieux expliquer notre démarche, laquelle n'est ni improvisée ni irrespectueuse des prérogatives du Parlement. Le Gouvernement souhaite effectivement que nous soyons prêts en mai prochain, et nous le serons. C'est pourquoi il a engagé, dès l'été dernier, le travail de transposition qui n'avait pas été mené auparavant en raison, notamment, des échéances électorales du premier semestre 2017. Après réflexion, le Gouvernement a fait le choix d'un texte resserré qui ne remette pas sur la table l'ensemble de la loi de 1978, ce que le droit européen n'exige nullement. Il s'agit de répondre à une problématique légistique nouvelle et complexe : tirer les conséquences d'un règlement d'application directe et d'une directive, dont les dispositions doivent être transposées dans la loi, alors que ces deux instruments européens portent sur des questions souvent similaires et, dans tous les cas, intrinsèquement liées. Vous reconnaissez vous-même dans votre rapport, madame Joissains, cette complexité inévitable.

Il ne s'agit aucunement de modifier ou de remettre en cause les apports du travail parlementaire. Il s'agit, encore une fois, d'une simple codification de nature légistique : plus qu'un engagement, c'est une responsabilité que porte le Gouvernement au nom de la stabilité de notre droit. Vous l'avez tous compris en lisant ce texte, l'accessibilité et l'intelligibilité du droit requièrent une réécriture intégrale de la loi de 1978 pour lui faire retrouver son ambition originelle, celle d'être un véritable code de la protection des données personnelles des Français.

du RGPD, un troisième titre relatif à la directive et un quatrième titre visant les dispositifs hors du champ de l'Union européenne. Mes services se tiennent à votre disposition pour vous informer régulièrement de l'avancement du projet d'ordonnance,

et par les professionnels au service des citoyens, des entreprises, mais également à l'attention des collectivités territoriales. Je suis d'ailleurs persuadée que nos débats auront aussi cette vertu pédagogique et qu'ils permettront d'écarter les inquiétudes les plus vives qu'il est normal de ressentir à l'occasion d'un tel changement de paradigme. Pour conclure, je souhaite que chacun puisse mesurer la portée de cette réforme à l'aune non seulement du projet de loi qui vous est proposé, mais plus largement des textes mis en oeuvre par l'Union européenne. L'exercice de transcription du droit européen présente toujours un caractère un peu contraint. Mais le nouveau cadre adopté par l'Union pour la protection des données personnelles est une magnifique réussite pour l'Europe et pour les citoyens de l'Union européenne. La parole

C'est une grande loi, une loi visionnaire, et si ses dispositions ont dû être adaptées au fil de l'évolution rapide des technologies numériques et du développement de nouveaux modes de traitement des données personnelles, ses principes cardinaux sont restés d'airain : consentement éclairé, loyauté de la collecte des données personnelles, adéquation aux finalités de traitement. Les traitements de données ont changé d'échelle et se sont mondialisés avec l'apparition de véritables géants numériques américains et, désormais, chinois. Dans cette course constante que se livrent le droit et la technique, le législateur européen, après de longues et âpres négociations, a adopté un règlement général sur la protection des données largement inspiré de la loi de 1978 et des travaux de la commission des affaires européennes du Sénat, et de son rapporteur, Simon Sutour, notamment sur l'extraterritorialité, l'un des points phares du projet de loi. Ce règlement entrera en vigueur le 25 mai 2018. Assorti d'une directive relative au traitement de données personnelles en matière policière et pénale, il entend promouvoir l'émergence d'un modèle européen harmonisé et ambitieux de la protection des données à caractère personnel tout en favorisant la compétitivité des entreprises européennes sur la scène internationale. Nous ne pouvons évidemment que souscrire à cet objectif. Et l'actualité récente nous montre combien il était urgent d'agir. Laissant un grand nombre de marges de manoeuvre aux États membres pour adapter certaines de ses dispositions, voire pour y déroger, le règlement poursuit trois objectifs principaux. Premièrement, il vise à renforcer les droits des personnes physiques en créant notamment un droit à l'oubli un droit à la portabilité des données personnelles et en facilitant l'exercice de ces droits- actions par mandataire, actions collectives, droit à réparation du préjudice Deuxièmement, il responsabilise tous les acteurs traitant des données en graduant leurs obligations en fonction des risques pour la vie privée, en privilégiant le recours à des outils de droit souple et en mettant fin à l'essentiel des formalités administratives préalables au bénéfice d'une obligation de conformité du traitement dès sa conception, ce qui est un véritable progrès. Troisièmement, crédibiliser la régulation à la mesure des enjeux de souveraineté numérique : l'extraterritorialité est consacrée, les autorités européennes sont appelées à coopérer pour contrôler et sanctionner en cas de traitement de données transfrontalier. Ces sanctions sont enfin réellement dissuasives 10 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial, chiffres pouvant même doubler dans certains cas ... Je ne m'attarderai pas sur la directive, qui reprend l'essentiel des principes du règlement et qui est applicable à tout traitement de données à caractère personnel aux fins de prévention, de détection des infractions pénales, d'enquêtes, de poursuites ou d'exécution des sanctions pénales. Elle doit être transposée avant le 6 mai 2018. Le projet de loi qu'il nous revient d'examiner a donc pour but d'adapter la loi de 1978- choix très symbolique -au règlement général, de tirer parti des marges de manoeuvre nationales qu'il autorise et de transposer la directive sectorielle. À cette fin, les missions de la CNIL sont élargies et ses pouvoirs renforcés. Le traitement des données dites sensibles reste très encadré et des régimes spécifiques plus protecteurs conservant des formalités préalables restent prévus pour certains traitements, notamment ceux qui visent le numéro de sécurité sociale, des données biométriques ou génétiques, des condamnations pénales, des archives ou des données de santé. L'Assemblée nationale a étendu l'objet de l'action de groupe en matière de données personnelles à la réparation des dommages en vue d'obtenir la réparation des préjudices matériels. Concernant la protection spécifique des données des enfants, les députés ont abaissé de seize à quinze ans l'âge à partir duquel un mineur peut consentir seul au traitement de ses données personnelles. Certaines décisions administratives individuelles fondées sur des algorithmes sont autorisées. Les règles applicables au traitement de données à caractère personnel prévues par la directive sont transposées. Enfin, le fichier de traitement d'antécédents judiciaires, le TAJ, est sécurisé en réponse à une décision QPC du Conseil constitutionnel. La commission des lois du Sénat, tout en approuvant les grandes orientations du projet de loi, a voulu réparer- je dois le dire, madame la garde des sceaux -de nombreuses lacunes et rééquilibrer certains éléments du dispositif. La Commission nationale de l'informatique et des libertés et le Conseil d'État s'accordent à constater l'illisibilité du projet de loi, alors que le contenu du règlement et de la directive était connu depuis avril 2016. En premier lieu, notre commission a tenu à répondre aux attentes et aux vives inquiétudes des collectivités territoriales. Ce sont les grandes absentes du projet de loi. Elles sont pourtant, de la plus petite à la plus grande d'entre elles, toutes- absolument toutes -concernées par les dispositions du règlement fichier d'état civil, fichier des cantines scolaires, fichiers d'aide sociale, listes électorales, fiscalité locale, cadastre ... Elles sont responsables de nombreux traitements sur lesquels elles n'ont souvent pas prise, car découlant d'obligations légales. Sous la menace de sanctions pécuniaires de la CNIL et de recours en justice, elles devront assumer seules des coûts importants : nomination d'un délégué à la protection des données, adaptation de certains fichiers existants, renforcement de la sécurité en cas de données sensibles, réponse à l'exercice des nouveaux droits des particuliers Les discussions à l'Assemblée nationale n'ont- hélas ! -pas permis de corriger les lacunes initiales du texte, car si nos collègues députés sont restés attentifs, à juste titre, au sort des TPE et des PME, les collectivités territoriales ont été totalement absentes des débats. Face à cette situation inédite, le Sénat, chambre des libertés et des collectivités territoriales, s'est ému. Sa commission des lois s'est attachée à prévoir que la CNIL adapte les normes qu'elle édicte et les informations qu'elle diffuse aux besoins et aux moyens des collectivités, notamment des plus petites d'entre elles, à dégager de nouveaux moyens pour aider celles-ci à se conformer à leurs nouvelles obligations et à faciliter la mutualisation des services numériques entre collectivités, à réduire l'aléa financier qui pèse sur elles, en supprimant la faculté offerte à la CNIL de leur imposer des amendes administratives. Elle a également voulu rééquilibrer la procédure d'action de groupe en réparation des dommages. Sans la remettre en cause, car elle est importante pour les droits des citoyens, il nous faut entendre l'inquiétude des petits opérateurs : chacun s'accorde à dire qu'ils ne seront pas prêts pour appliquer le règlement européen dès le 25 mai 2018-

Dans le but d'apporter des solutions concrètes à ces problèmes spécifiques, la commission des lois a proposé de différer de deux ans l'entrée en vigueur de l'action de groupe en réparation des dommages et d'imposer, de même qu'en droit de la consommation ou de l'environnement, un agrément préalable des associations de protection de la vie privée pour introduire une action de groupe.

conformément au droit commun européen et dans l'attente de travaux plus approfondis de nature à dégager de véritables critères d'évaluation, ainsi qu'un régime d'accompagnement adapté. La présidente de la commission de la culture, Catherine Morin-Desailly, y travaille assidûment. La commission a également veillé à encadrer strictement l'usage des algorithmes par l'administration dans la prise de décisions individuelles. Elle a tenu à renforcer les garanties de transparence en la matière, notamment pour les inscriptions à l'université qui ne doivent pas constituer une exception au droit à l'information dû à tout un chacun. La commission a rétabli l'autorisation préalable des traitements de données portant sur les infractions, condamnations et mesures de sûreté. Elle a précisé les conditions d'extension de la liste des personnes autorisées à mettre en oeuvre ces fichiers, ainsi que le cadre juridique de la mise à disposition des décisions de justice en, et ce ce afin de prévenir tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes, mais aussi de préserver l'indépendance et la liberté d'appréciation de la justice. Souhaitant porter le débat en séance et innover en la matière, elle a adopté un amendement visant à s'assurer que les utilisateurs de terminaux électroniques ne soient pas victimes d'un choix par défaut et qu'ils aient la possibilité d'installer sur leur terminal d'autres moteurs de recherche que celui qui est imposé par le fabriquant, et notamment des moteurs de recherche respectueux de la vie privée. Enfin, la commission des lois a supprimé l'habilitation demandée par le Gouvernement pour procéder par ordonnance aux corrections des très nombreuses incohérences subsistant entre le droit français et le droit européen. Regrettant le manque d'anticipation du Gouvernement, qui a témoigné, je dois le dire, d'une grande désinvolture vis-à-vis du Parlement et d'une ignorance difficilement compréhensible des collectivités,

Si nous partageons pleinement l'esprit et les objectifs des textes européens et la volonté de maintien de la loi de 1978 dans le projet de loi, je ne saurais conclure sans insister sur l'importance des nouvelles missions attribuées à la CNIL. cette dernière que reposent tout le nouvel édifice de protection des droits et la responsabilité d'accompagner les acteurs économiques et les élus locaux. Je souhaite vous interroger solennellement, madame la garde des sceaux, sur le grave problème que va poser l'insuffisance des moyens L'autorité, déjà très sollicitée, n'a pas, en l'état, les capacités matérielles et humaines de faire face à sa nouvelle charge de travail. Les quelques mesures que nous avons proposées pour faciliter son organisation interne n'y suffiront pas. Que pouvez-vous nous dire, à ce stade, des engagements budgétaires et humains qui devront nécessairement être pris par le Gouvernement ? Il y va de la réussite même de cette ambitieuse réforme de la protection des données. La parole Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le 21 février dernier, la conférence des présidents a décidé de confier à la commission des affaires européennes, à titre expérimental, une mission de veille sur l'intégration des normes européennes en droit interne. C'est dans cette optique que la commission des affaires européennes a examiné le présent projet de loi et formulé un ensemble d'observations. Le règlement européen sur la protection des données personnelles s'appliquera de plein droit à compter du 25 mai prochain.

Cette situation illustre, si besoin est, la nécessité d'une participation active du Parlement, et singulièrement du Sénat, représentant constitutionnel des collectivités locales, à l'élaboration des textes européens. Il nous faut, en particulier, pouvoir anticiper et attirer l'attention du Gouvernement sur les conséquences concrètes de ceux-ci. La discussion du règlement général sur la protection des données personnelles a fait l'objet d'un suivi attentif de la commission des affaires européennes. J'ai notamment déposé et rapporté, en son nom et au nom de la commission des lois, deux propositions de résolution européenne et produit un avis motivé. Les résolutions du Sénat demandaient que des dispositions nationales plus protectrices puissent être conservées et que toute personne résidant en France soit en droit de saisir la CNIL, même si le siège de l'entreprise traitant ses données est situé dans un autre État membre. Première observation : le règlement général sur la protection des données reprend les deux éléments que le Sénat avait mis en avant. L'autorité de contrôle compétente est bien celle de la résidence du demandeur.

de limiter les droits des personnes pour des motifs stricts de sécurité publique. Le projet de loi exploite certaines de ces marges de manoeuvre, en particulier pour maintenir, tout en les révisant, des régimes spéciaux

La commission des affaires européennes estime que cette question doit faire l'objet d'une approche mesurée. Le texte adopté par la commission des lois va tout à fait dans ce sens. Troisième observation : l'extension Troisième observation : l'extension de l'action de groupe à la réparation pécuniaire, introduite par l'Assemblée nationale, n'est pas prévue par le règlement général, mais il s'agit d'une faculté ouverte par le droit européen pour d'autres actions de groupe, raison pour laquelle la commission des affaires européennes recommande qu'elle soit envisagée à l'échelon européen et assortie de règles renforcées d'enregistrement des associations. Il s'agit, là encore, d'une approche partagée par la commission des lois. Quatrième observation : la nécessité de s'assurer de la protection effective des données et des droits des personnes en cas de transfert vers des pays tiers. Dans son premier rapport d'application de l'accord sur le bouclier de protection conclu entre l'Union européenne et les États-Unis, la Commission européenne estime la Commission européenne estime que la mise en oeuvre de cet accord doit être améliorée, en particulier la vérification de la conformité des entreprises qui se sont autocertifiées. Il conviendra donc de suivre attentivement cette question.

Il est donc à tout le moins indispensable d'organiser un accompagnement adapté, voire très adapté, comme le prévoit la commission des lois, et d'y associer pleinement la CNIL, dont les moyens, notamment techniques, doivent être rapidement renforcés. Le Sénat et sa commission des affaires européennes entendent être vigilants quant au suivi de l'élaboration et de la mise en oeuvre des textes européens.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs décennies, l'insécurité numérique s'est développée à une vitesse folle, faute de contre-pouvoir souverain et protecteur. Nous assistons, impuissants, au pillage de nos données personnelles par les géants américains de l'Internet, les Vador du numérique, les fameux GAFA- Google, Apple, Facebook et Amazon, publicité non rémunérée ... Pillage des données personnelles des individus, mais aussi de nos entreprises et même de nos États. Ces grandes firmes se les approprient, les stockent, les utilisent gratuitement et les monétisent. Toute notre vie est observée puis orientée. Le du roman de George Orwell est devenu réalité : souriez, vous êtes scannés. Détendez-vous, on pense pour vous. Vos goûts, vos désirs, vos opinions sont épiés, disséqués, analysés pour être influencés. L'oeil du cyclone ne vous laissera pas faire un pas seul. Et son immense puissance, c'est de vous faire croire que Quels que soient nos choix, nos achats, notre géolocalisation, le croisement des données réalisé par l'intelligence artificielle permet aux grosses firmes de nous connaître intimement et d'utiliser nos données, sans notre accord, pour générer des milliards et encore des milliards de profits. Dans cette guerre du numérique, ces utilisations à des fins commerciales portent atteinte à la liberté des individus, mais c'est encore plus grave quand il s'agit des données de nos entreprises stratégiques ou de nos administrations, livrées à ces multinationales.

Pourquoi sommes-nous contraints d'être dépendants de logiciels américains et bientôt chinois, qui espionnent ainsi nos activités économiques et personnelles ? Il est grand temps de nous saisir de ce dossier, en prenant immédiatement les mesures qui s'imposent : mieux informer les utilisateurs français sur la récupération de leurs données personnelles, dès lors qu'ils valident les conditions générales d'utilisation harmoniser au niveau national le droit numérique par la création d'un code incluant à la fois la législation européenne, la législation nationale et les normes existantes ; instaurer l'obligation de stocker les données personnelles dans des serveurs en France, avec interdiction de les transférer développer les solutions de logiciels libres, notamment dans les administrations, les universités et les écoles, tout en encourageant leur utilisation par le grand public ; ouvrir, à l'échelon européen, avec tous les pays qui le souhaitent, un projet de coopération en matière de numérique visant à préserver la sécurité et la souveraineté de nos États et la liberté de nos citoyens. Nous avons besoin d'une agence européenne, qui développerait, comme Airbus pour l'aéronautique, des champions français et européens du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Je salue l'avancée permise par ce texte, qui permettra une meilleure protection des Français. Il est un levier pour la mise en place de bonnes pratiques dans les entreprises, notamment sur les questions de sécurité. La commission des lois a porté un regard attentif aux petites entreprises et aux collectivités territoriales, ce qui est louable. Ne l'oublions pas, dans le domaine numérique comme dans tous les autres, ce qui prévaut, c'est avant tout notre souveraineté.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, si le texte que nous examinons aujourd'hui a pour principal objet d'assurer la conformité de notre droit national avec le droit européen, il soulève toutefois plusieurs questions qui méritent d'être plus longuement discutées au sein de notre assemblée. L'adoption en 2016 du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, le RGPD, constitue un progrès indéniable sur le plan européen. Il s'agit également d'une victoire diplomatique française, ce règlement visant à faire converger les droits des États membres vers des standards plus protecteurs des données personnelles, proches des standards français. Il est vrai que, depuis la loi du 6 janvier 1978, notre pays a joué un rôle précurseur en la matière. Ce règlement européen est également réaliste. Il prend acte du formidable développement des données personnelles en circulation qui constituent aujourd'hui la matière première de nombreuses entreprises, en transformant la logique d'autorisation en logique de responsabilisation des acteurs du marché. Il revient désormais à ces derniers de s'assurer que leurs traitements des données sont effectués en conformité avec les règles applicables en matière de collecte. Ces impératifs du RGPD concernant la licéité de la collecte, le consentement des individus dont les données sont collectées, ou encore la finalité du traitement des données s'imposent donc à tous, acteurs privés, mais également acteurs publics ... Je pense évidemment à nos collectivités territoriales Au sein de toutes ces structures, en particulier les plus petites et les moins bien informées, l'application du RGPD est un défi, un « changement de paradigme », comme l'ont évoqué certains, qui mériterait un meilleur accompagnement par l'État.

avec la nomination d'un délégué à la protection des données et la mise en place d'un meilleur ciblage du traitement concernant les données sensibles et les mineurs, a bouleversé les habitudes. Elle a également nécessité un ciblage des hébergements des données personnelles sous-traitées à l'extérieur du réseau du département, la mise en oeuvre d'un registre des traitements priorisé sur les données sensibles, enfin, une communication à destination des usagers, notamment au vu des obligations en termes de consentement. Ainsi, c'est toute une organisation, avec des processus et des mesures dont je vous épargnerai le nom, qui a dû être mise en place pour assurer la conformité avec ce règlement et une réelle protection des données de nos concitoyens. s'agit enfin d'un énorme travail à destination des agents, notamment en termes de formation sur le traitement des données sensibles et, surtout, sur la conservation des données de manière générale. D'une part, le coût global de ces transformations est largement sous-estimé. D'autre part, l'absence de prise en compte des difficultés que rencontrent de nombreuses collectivités territoriales donne lieu à une protection inégale des données personnelles de nos concitoyens, selon qu'ils sont domiciliés dans une collectivité respectueuse ou non du RGPD. C'est pourquoi je tiens à saluer le travail important effectué par notre collègue Sophie Joissains, qui a procédé à un grand nombre de modifications en faveur des collectivités territoriales, mais également des petites entreprises. Malgré les difficultés matérielles de mise en oeuvre, je souhaite insister sur plusieurs dispositions importantes du projet de loi qui permettront une amélioration de la protection de nos données personnelles. Je pense, par exemple, à la facilitation des actions en justice, notamment à la création d'une action de groupe. Je pense aussi à la possibilité donnée à la CNIL de saisir le Conseil d'État pour qu'il puisse ordonner la suspension du transfert des données en cause, dans l'attente d'une décision définitive de la Cour de justice de l'Union européenne. Ces dispositions contribueront effectivement à la protection des données personnelles des Français. La question de la fixation d'un âge légal de consentement au partage de données personnelles devrait également donner lieu à de nombreux débats. Sur ce point, deux visions se dégagent, certains considérant que cet âge devrait être le même que celui de l'émancipation, d'autres souhaitant responsabiliser progressivement les adolescents. À nos yeux, cette question devrait être abordée dans le cadre d'une approche globale de l'accès à la majorité. Après la phase de découverte des possibilités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous entrons dans une phase de prudence et de prise de conscience de l'impact potentiel de l'utilisation de ces technologies sur nos libertés publiques et individuelles. Nous regrettons donc que ce projet de loi ne réponde pas à l'ensemble des préoccupations des Français. La question du consentement à l'utilisation des données personnelles est légitime, et reviendra sûrement au cours de nos prochains débats. Il convient de réfléchir au financement des services proposés par des sites internet, lesquels font valoir que l'exploitation des données personnelles à des fins de publicité est la contrepartie de la gratuité de leurs services. La création de droits sur les données personnelles remettrait en cause ce modèle de financement. Un tel sujet mérite d'être débattu, dès lors que les Français attendent une plus grande traçabilité des informations les concernant. Il en va de même s'agissant des algorithmes utilisés par l'administration, à la suite des vives critiques qui se sont élevées contre le traitement automatisé du système admission post-bac. La solution proposée par Mme la rapporteur est plus satisfaisante que la version issue des travaux de l'Assemblée nationale, mais nous considérons que le dispositif pourrait encore être amélioré.

Enfin, l'existence de marges de manoeuvre autorisées par le règlement européen nous inquiète, dès lors que celles-ci pourraient encourager la localisation de sous-traitants des responsables de données personnelles dans les États membres les moins protecteurs. C'est pourquoi nous avons proposé plusieurs amendements destinés à alerter le Gouvernement sur les risques que cela pourrait comporter pour nos concitoyens et sur la situation difficile dans laquelle se trouveront nos entreprises de traitement de données personnelles, très protectrices en la matière, face à leurs concurrents localisés dans les États offrant moins de

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame la rapporteur, mes chers collègues, alors que le règlement européen relatif aux données personnelles doit entrer en vigueur à compter du 6 mai 2018, l'adoption du présent projet de loi revêt un caractère incontournable. indépendamment de cette obligation liée à nos engagements européens, l'adaptation de notre législation au formidable défi soulevé par les questions liées aux n'en était pas moins urgente. pas plus que les géants de l'Internet, les pirates ou profiteurs de tout poil n'attendront pas l'adaptation de notre législation pour exploiter sans vergogne les données personnelles de nos concitoyens. Pour organiser un dispositif de sécurité efficace, l'Union européenne est une chance pour la France, car elle constitue l'échelon le plus pertinent. Comme l'ont souligné Mme la rapporteur et M. Sutour, le RGPD permet aux États membres d'harmoniser leurs pratiques, en prenant exemple sur ce qui fonctionne chez leurs voisins, ce qui leur laisse une marge très appréciable pour mener leurs propres politiques d'adaptation. Ils pourront d'ailleurs s'inspirer de la France, précurseur en matière de protection des données, puisque nous fêtons cette année les quarante années d'existence de la CNIL, d'ailleurs présidée en son temps par notre ancien collègue Alex Türk. Les données personnelles touchent donc à la vie privée, à la santé, à nos comportements, par le biais de photos ou d'informations ... bref, à l'intime. Il me semble que c'est déjà se faire une certaine idée de l'homme et de l'État de droit que de considérer que le citoyen ne peut être dépossédé de cette intimité. En affirmant son refus de laisser à des tiers une emprise sur nos existences, le Sénat remplit pleinement sa vocation de défenseur des libertés individuelles. Au travers de ce projet de loi, c'est aussi l'occasion d'affirmer une certaine conception de la démocratie, d'autant que les révélations faites par deux journaux américains nous dessinent un horizon particulièrement sombre en la matière. En effet, si elle était confirmée, la captation par l'entreprise prétendument académiques, de données recueillies sur Facebook émanant de 30 à 50 millions de comptes à des fins de profilage politique pour influencer le vote lors de la dernière élection présidentielle américaine montre l'acuité de la menace.

Mais l'existence de ces données personnelles peut aussi être, à condition de voir leur utilisation très solidement encadrée, une opportunité économique, et même une formidable chance pour la recherche médicale. Sur le projet de loi tel qu'il nous a été transmis par l'Assemblée nationale, le travail effectué par nos rapporteurs a été remarquable. Je tiens notamment à saluer les nombreux apports que Sophie Joissains a fait intégrer dans le texte adopté par la commission des lois. Je ne reviendrai pas sur les nombreuses dispositions que comporte le texte du Gouvernement et qui viennent d'être amplement détaillées, mais je souhaite m'arrêter sur un point sur lequel vous avez, madame la rapporteur, apporté une avancée décisive : il concerne les collectivités locales. En effet, il s'agissait là du parent pauvre du texte : rien sur l'état civil, les cadastres, les fichiers des centres communaux d'action sociale ou les listes électorales. Parce qu'elles sont au centre de la vie quotidienne de nos concitoyens, les collectivités sont les premières concernées par l'utilisation de leurs données personnelles. Mais en imposant à la CNIL d'adapter les normes à leurs besoins, vous avez rendu possible ce qui, avec les moyens matériels et humains actuels, ne l'aurait sans doute pas été. Parmi les avancées déterminantes intégrées par la commission des lois, je veux citer aussi la mutualisation des services supports offerts par les syndicats mixtes au bénéfice des communes et des intercommunalités ; la création des dotations communales et intercommunales pour la protection des données personnelles point essentiel à l'heure de la baisse des dotations - sur les recettes de l'État ; l'exonération des collectivités des amendes et astreintes administratives en cas de sanction. En comblant ces lacunes, vous avez rappelé, madame la rapporteur, que le Sénat est plus que jamais l'assemblée des collectivités territoriales et celle des solutions pratiques. Voilà qui devrait faire réfléchir avant d'affaiblir le bicamérisme, lequel fait la richesse de nos institutions.

aux TPE-PME de s'organiser pour se conformer à leurs nouvelles obligations. Ne pas laisser aux responsables de traitement ce laps de temps aurait été parfaitement déloyal au regard de leurs moyens, et aurait eu pour conséquence de les exposer directement à des actions de groupe. En effet, les nouvelles règles dont nous débattons aujourd'hui sont certes salutaires, mais aussi particulièrement lourdes à mettre en place. Peu nombreuses sont les PME qui disposent dans l'immédiat de l'ingénierie nécessaire. Alors que Alors que nous venons d'adopter cet après-midi le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance qui admet le droit à l'erreur, il serait profondément inéquitable et choquant que l'administration soit plus prompte à sanctionner des PME que les GAFA, dont on connaît les ressources juridiques pour faire durer des procédures-fleuves. Certes, on ne peut que déplorer que les précédents gouvernements n'aient pas pris la mesure du travail législatif à accomplir. Mais nous sommes nombreux à regretter, sur les travées de la Haute Assemblée, que le Gouvernement n'ait pas réalisé en amont le travail qui devait être mené auprès des PME et des collectivités locales. Il s'appuie à présent sur ses propres manquements pour justifier le recours aux ordonnances initialement inscrit à l'article 20 du texte transmis par l'Assemblée nationale, ce qui constitue une nouvelle illustration de la mise à distance d'un parlement amputé de ses prérogatives. Pour recodifier la loi Informatique et libertés de 1978, le Gouvernement souhaite aujourd'hui légiférer dans l'urgence par ordonnances, alors que la publication, en et de la directive lui laissait amplement le temps d'agir. Permettez-moi donc de souscrire au signal que vous avez envoyé, madame la rapporteur, à l'heure où d'aucuns souhaitent réformer le Parlement pour pallier son supposé manque d'efficacité. Je conclurai en formulant le voeu que ce texte soit interprété par le Gouvernement et par la CNIL comme un outil salutaire visant à protéger les citoyens, grâce à l'adoption d'armes efficaces contre les mastodontes de l'internet, et non comme un nouveau monstre juridique assommant nos collectivités locales et nos PME. Très bien

de « malaisé ». La grande disparité des régimes de protection au sein de l'Union, l'attention aiguisée de certains États, particulièrement la France, sur les données dites sensibles, les enjeux de souveraineté et les demandes de simplification des entreprises

La Chancellerie a donc déployé des efforts considérables pour mener à bien cette transposition extrêmement ardue dans des délais très courts.

consciente de l'inquiétude que peut susciter un nouveau cadre législatif, a proposé une série d'amendements. En effet, seuls 2 % de nos communes ont pris conscience du problème et commencé à engager un certain nombre de procédures,

à l'action de la CNIL, leurs besoins spécifiques, à les exonérer, au même titre que l'État, en raison de leurs prérogatives de puissance publique, de l'amende administrative et de l'astreinte, à faciliter la mutualisation des services numériques entre collectivités, ou encore

les difficultés rencontrées par nos territoires, notamment l'absence de prise en compte de ce sujet par les collectivités, principalement les communes. Nous ne pouvons que nous féliciter que le Gouvernement

la suppression pour les collectivités locales de l'amende administrative et de l'astreinte prévue à l'article 6 du texte. Je veux également évoquer l'action de groupe, introduite en France très tardivement, en 2014. Notre collègue députée Paula Forteza a souhaité en étendre le champ en constatation d'un manquement du responsable de traitement ou de son sous-traitant.

le texte issu des travaux de la commission reporte à deux ans l'entrée en vigueur de ce recours, ce qui permet aux acteurs concernés, particulièrement aux collectivités locales, de s'adapter. Enfin, comme cela a pu être mentionné, la France avait été pionnière en se dotant d'une législation globale de protection des données à caractère personnel, avec la loi du 6 janvier 1978, mais également d'une autorité de contrôle, la CNIL. Le Gouvernement a fait le choix de maintenir la loi de 1978, car, au-delà de sa portée symbolique, elle n'était pas visée dans sa totalité par les nouvelles normes européennes, ce qui permet au Parlement de procéder à l'examen d'un texte ne contenant que les dispositions affectées par le droit européen, plutôt qu'à une remise en question des dispositions existantes et satisfaisantes de la loi de 1978, telle que modifiée. Les délais l'exigeaient sans doute également. Le Gouvernement a donc sollicité du Parlement une habilitation pour codifier par la suite les modifications apportées à notre droit par le projet de loi que nous examinons, afin d'offrir un cadre juridique lisible aux citoyens et aux acteurs économiques. La commission des lois a relevé une certaine illisibilité Il serait en conséquence paradoxal que le Sénat s'oppose à l'habilitation par voie d'amendement. Le Gouvernement s'est engagé à respecter le texte voté par les assemblées, l'habilitation proposée dans le texte initial fixant clairement un cadre. Les dispositions de fond ont été débattues à l'Assemblée nationale, elles le sont aujourd'hui au Sénat. Le temps parlementaire est précieux, cela est souvent relevé dans cette enceinte. Finalement, l'habilitation à légiférer par ordonnance permet de le respecter.

le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui a pour objet de mettre la loi de 1978 en conformité avec le droit de l'Union européenne. Il transpose le règlement règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la directive 2016/680 par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. Avant de traiter du fond, permettez-moi, mes chers collègues, quelques remarques liminaires sur la forme. Ces deux instruments juridiques européens ont été adoptés en 2016, leur entrée en vigueur étant Cette date était connue de tous, tout comme les modifications de notre droit qu'ils rendaient nécessaires. Aussi regrettons-nous que, sur un sujet d'une telle importance, le Gouvernement ait tant tardé à déposer ce projet de loi et qu'il ait, une fois de plus, déclenché la procédure accélérée. Il propose en outre, par le biais de l'article 20, prétendument pour respecter les délais, de réformer la loi de 1978 par voie d'ordonnance.

dans le cadre de la réforme des institutions, ne s'agit-il pas plutôt d'une illustration supplémentaire du profond mépris du Gouvernement à l'endroit du Parlement ? Cela dit, venons-en, mes chers collègues, au fond du texte qui nous réunit aujourd'hui. Il contient des avancées fondamentales pour la protection des données personnelles de nos concitoyens. Le temps qui m'est imparti ne me permettant pas de commenter chacune des dispositions de ce projet de loi dense et technique, je ne prendrai que deux exemples. j'évoquerai l'aménagement et le renforcement des pouvoirs et des compétences de la CNIL, qui se voit désigner autorité nationale de contrôle chargée de veiller à l'application du règlement et de la directive. de loi prévoit la réduction des formalités préalables pour la mise en oeuvre des traitements comportant le moins de risques

En contrepartie, la CNIL voit ses pouvoirs de contrôle et de sanction renforcés, avec la possibilité d'infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'organisme concerné. Nous nous félicitons, bien sûr, de ces évolutions, mais nous partageons l'inquiétude de la CNIL, qui alerte, depuis plusieurs mois, sur un défaut de moyens matériels et humains qui ne lui permettra pas d'exercer efficacement ses nouvelles missions. C'est bien d'être approuvée ! Cela ne m'arrive pas souvent ! Deuxièmement, je rappellerai le renforcement, en matière pénale, des droits des personnes, puisque le texte crée un droit à l'information et prévoit l'exercice direct de droits tels que les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données, donc le droit à l'oubli. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste se réjouit de l'adoption de ces mesures plus protectrices. Finalement, ce n'est pas tant ce que le présent projet de loi contient qui appelle, de la part du groupe CRCE, des commentaires, que ce qu'il ne contient pas. Nous considérons en effet que les prérogatives accordées aux services de renseignement français par la loi Renseignement de 2015 devraient également être mises en conformité avec les dispositions de la directive, et donc introduites dans le texte dont nous débattons aujourd'hui. Tel n'est toutefois pas le cas. Ce projet de loi, porté par un gouvernement qui ne souhaite en aucun cas rouvrir le débat sur ce sujet, ne contient aucune disposition de nature à mettre le droit français en conformité avec le droit de l'Union européenne en la matière et à respecter, enfin, les droits fondamentaux de nos concitoyens, bafoués sur nombre de points par la loi Renseignement, votée sous le gouvernement précédent, je le précise. Rappelons que cette même loi Renseignement a déjà été censurée trois fois par le Conseil constitutionnel, et que d'autres recours et questions prioritaires C'est donc avec le sentiment d'une occasion manquée que le groupe CRCE s'abstiendra sur ce texte qui, s'il constitue, sans aucun doute, un pas de plus dans la construction du droit commun européen, aurait pu être plus ambitieux et garantir à l'ensemble de nos concitoyens le respect effectif de leurs libertés individuelles. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'objet du projet de loi relatif à la protection des données personnelles est d'adapter notre droit au « paquet européen de protection des données personnelles qui se compose d'un règlement général sur cette protection et d'une directive spécifique aux traitements mis en oeuvre en matière policière et judiciaire. Les délais sont très limités : nous devons avoir transposé la directive avant le 6 mai prochain, et le règlement doit être directement applicable à partir du 25 mai Concernant en premier lieu le règlement européen, celui-ci doit constituer le nouveau cadre de la protection des données personnelles des Européens tout en protégeant la compétitivité des entreprises européennes. son application est atténuée par l'existence de 56 marges de manoeuvre, qui sont autant d'options facultatives ou de dérogations que les États peuvent introduire dans leur droit national. poursuivent principalement trois objectifs. Il s'agit, premier objectif, de renforcer les droits des personnes dont les données sont utilisées : le règlement réaffirme les droits des personnes, introduit de nouveaux droits mieux adaptés à l'évolution des technologies numériques et facilite l'exercice de ces droits par des actions par mandataire, voire par des actions collectives, tout en promouvant le droit à réparation du préjudice subi. Le deuxième objectif du règlement est de mieux graduer les obligations des acteurs en fonction des risques pour la vie privée. Le troisième objectif est de doter les régulateurs de pouvoirs à la mesure des enjeux de souveraineté numérique. Le champ d'application territorial et matériel du droit européen est considérablement élargi : le règlement doit non seulement être appliqué lorsque le responsable de traitement est établi sur le territoire de l'Union européenne, mais il a également vocation à s'appliquer hors de l'Union, dès lors qu'un résident européen est visé par un traitement de données. Les règles de transfert des données personnelles hors de l'Union européenne sont précisées et la coopération entre régulateurs en cas de transferts transfrontaliers est considérablement renforcée. en cas de manquement, des amendes désormais dissuasives, jusqu'à 10 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial. En second lieu, concernant la directive, celle-ci reprend l'essentiel des principes du règlement et est applicable à tout traitement de données à caractère personnel aux fins de prévention, de détection des infractions pénales, d'enquêtes, de poursuites ou d'exécution de sanctions pénales. Lors de l'examen du texte en commission des lois, un certain nombre d'améliorations ont été apportées. Ainsi, dans le domaine de la justice, la commission a rétabli l'autorisation préalable des traitements de données portant sur les infractions, condamnations et mesures de sûreté, précisé les conditions d'extension de la liste des personnes autorisées à mettre en oeuvre ces fichiers, ainsi que le cadre juridique de la mise à disposition des décisions de justice, afin de prévenir tout risque d'atteinte tant à la vie privée des personnes qu'à l'indépendance de la justice. La commission des lois a aussi strictement encadré l'usage des algorithmes par l'administration lorsque cette dernière prend des décisions individuelles. Elle a en outre renforcé les garanties de transparence en la matière, par exemple pour les inscriptions à l'université. Je voudrais saluer ici le travail accompli par la rapporteur de la commission des lois, qui a répondu aux attentes et aux vives inquiétudes des collectivités territoriales. sous la menace de sanctions pécuniaires, les collectivités devront assumer seules des coûts importants relatifs, entre autres, au renforcement de la sécurité en cas de données sensibles, à la nomination d'un délégué à la protection des données ou encore à l'adaptation de certains fichiers existants. Face à cette situation, la commission des lois s'est attachée à dégager de nouveaux moyens financiers pour les aider à se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions, en fléchant le produit des amendes et astreintes prononcées par la CNIL à leur intention et en créant une dotation communale et intercommunale pour la protection des données personnelles. La commission des lois a également facilité la mutualisation des services numériques entre collectivités territoriales. Afin de réduire l'aléa financier pesant sur ces dernières, elle a supprimé la faculté pour la CNIL de leur imposer des amendes administratives et a reporté de deux ans l'entrée en vigueur de l'action de groupe en réparation de préjudices en matière de données personnelles. Enfin, la commission des lois a encouragé la diffusion d'informations et l'édiction de normes de droit souple par la CNIL, adaptées aux besoins et aux moyens des collectivités territoriales comme des TPE et PME. Madame la ministre, mes chers collègues, le sort réservé aux collectivités territoriales nous inquiète tout particulièrement, car le règlement s'imposera à elles aussi dès le mois de mai. ! Je me réjouis donc que la commission des lois, par l'entremise de son rapporteur, dont je salue ici le travail très efficace, ait dégagé deux pistes très importantes : exonérer les collectivités de certaines sanctions et les aider à financer et à gérer les outils devenus nécessaires. Aussi, la commission des lois ayant été attentive aux fortes préoccupations des collectivités territoriales et ayant renforcé par ailleurs les garanties en faveur des libertés individuelles, voterai-je, et mon groupe avec moi, pour l'adoption de ce projet de loi.

contrairement aux apparences, le texte que le Sénat est amené à examiner aujourd'hui n'est pas qu'un texte technique, qui n'intéresserait par définition que ceux d'entre nous qui attachent de l'importance aux questions numériques.

ans après l'adoption de la loi Informatique et libertés, en 1978, notre pays défend son modèle et réinvente, dans un cadre européen affirmé, la protection des données personnelles en l'adaptant aux temps nouveaux. et libertés ait été maintes fois modifiée, au gré des évolutions techniques et sociétales, ses grands principes sont confortés. Je m'en félicite d'autant plus que j'ai la chance de pouvoir siéger au sein de la CNIL, où je représente le Sénat avec notre collègue Sylvie Robert.

Parce qu'elles « appartiennent » à chaque citoyen, parce qu'elles nous caractérisent, parce que, massifiées, reliées, moulinées par un algorithme, elles peuvent avoir un intérêt majeur pour tout un tas d'acteurs, économiques ou autres,

On estime que cette société aurait « aspiré », puis conservé, les données personnelles de dizaines de millions d'électeurs américains dans le but de les cibler au profit de la campagne de Donald Trump. Cette collecte s'est faite, dans la majorité des cas, sans le consentement des utilisateurs du réseau social Facebook. N'en déplaise, alors, aux Cassandre, aux chantres de la dérégulation à tous crins ou à ceux que notre ancien collègue sénateur et ancien président de la CNIL, Alex Türk, qualifiait de tenants du « rien à cacher, rien à me reprocher », notre législation constitue un véritable bouclier protecteur, que ce texte ne vient que renforcer. Qu'il s'agisse des libertés publiques, de la sécurité et de la souveraineté, la question des données personnelles constitue bien la nouvelle frontière du monde nouveau. Le changement de paradigme que vous avez évoqué, madame la ministre, réside dans la responsabilisation des acteurs eux-mêmes, qu'ils soient publics ou privés.

une question subséquente se pose néanmoins- je remercie notre collègue Esther Benbassa de l'avoir dit aussi clairement - : celle des moyens de cette autorité administrative indépendante. Tout le monde conviendra que, si le rôle de la CNIL change de nature, celle-ci devra recevoir du budget de l'État les moyens d'accomplir ses missions, au même niveau au moins que dans les grandes nations européennes qui nous entourent. Le monde qui vient n'est pas un monde anxiogène, pas plus que ne l'était le monde de 1978. Et c'est dans cet esprit positif que le groupe Union Centriste aborde ce texte, en soutenant les améliorations sur le fond apportées par la commission des lois sur les propositions de Mme le rapporteur et de certains de nos collègues. À ce titre, je souhaiterais tout particulièrement insister sur la question des entreprises,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quand le législateur s'intéresse aux questions d'innovation et aux questions numériques, il est confronté à une difficulté majeure : l'évolution de la société qu'il essaie de réguler est-elle achevée ? Rappelez-vous des premières réactions apparues lorsque certains ont voulu porter le fer contre Airbnb : ils ont été accusés d'aller contre la disruption technologique, le progrès, l'ordre numérique des choses. Puis le berceau même d'Airbnb, la ville de San Francisco, a engagé un mouvement de régulation du site. Aujourd'hui, le mouvement est quasi global : à Londres, à Barcelone, à San Francisco ou à Paris, les pouvoirs publics cherchent à contrôler la plateforme, avec le soutien d'une opinion qui ne percevait pas encore, il y a quelques années, les effets pervers d'Airbnb sur l'environnement urbain et sur l'hôtellerie. Qu'en est-il des mesures qui nous sont proposées aujourd'hui ? Bien sûr, la vision des enjeux relatifs à la protection des données personnelles contenue dans le projet de loi que nous étudions a déjà quelques années. Elle est directement issue de débats européens que l'on peut situer entre 2014 et 2016. Évidemment, le concept de données personnelles n'a pas énormément évolué depuis cette période. Mais peut-être en va-t-il différemment de notre perception ? En 2014, je pouvais imaginer que mes données personnelles échappent à mon contrôle total. Le principal enjeu était sans doute le déréférencement de données personnelles traînant sur internet. Les GAFA, à cette époque, étaient perçus comme des champions enviables, qui pouvaient chercher, de temps à autre, à frauder le fisc. Mark Zuckerberg a été élu homme de l'année, en 2010, Aujourd'hui, nous savons que des soldats français voient leur position confidentielle divulguée à cause de leur utilisation d'objets connectés ; nous savons que Donald Trump a utilisé les services d'une société qui a volé les données personnelles de millions d'Américains ; nous savons que des puissances étrangères n'hésitent pas à profiler des millions d'utilisateurs et à créer de faux profils pour influencer des élections dans d'autres pays. Nous savons aussi que le pays de naissance des GAFA commence à envisager de contrôler de manière beaucoup plus forte ses propres licornes numériques, de peur qu'elles ne deviennent incontrôlables. À l'aune de ces quelques constats, je crois pouvoir affirmer que ce texte va dans le bon sens, même s'il ne règle pas l'ensemble des problématiques fluctuantes liées aux données personnelles. Le débat, déjà riche à l'Assemblée nationale, a également été très intéressant, ici, en commission des lois, grâce au travail de notre rapporteur Sophie Joissains. Je pense d'abord aux aménagements proposés pour permettre aux collectivités locales- c'est le rôle du Sénat -de se mettre en accord avec les nouvelles dispositions relatives à la protection des données personnelles. Ces dérogations déplairont sans doute aux bons élèves qui ont déjà oeuvré pour se mettre en conformité avec leurs obligations en amont des échéances légales. Mais elles permettront au peloton des nombreuses collectivités et des entreprises concernées dans notre pays de suivre le mouvement. Ces dérogations permettront aussi que se déploie l'offre de services en direction des collectivités locales. Je pense plus particulièrement, ici, aux nécessaires mutualisations proposées aux 90 % de petites collectivités qui sont souvent encore ignorantes de leurs obligations en la matière. confié, par exemple, aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, dont certains se sont déjà positionnés sur ces services. Le groupe socialiste et républicain a déposé une vingtaine d'amendements sur ce texte. Leur examen nous permettra, aujourd'hui et demain, de nous attarder sur le secret médical, de réfléchir à la sécurité des données intéressant la sûreté de l'État, d'envisager la suppression de l'agrément de l'autorité administrative auquel est aujourd'hui soumise toute action de groupe en matière de données personnelles, ou encore de limiter plus étroitement le recours aux algorithmes. Je tiens par ailleurs à exprimer mon soutien aux initiatives visant à garantir que des contrats ne s'opposent plus à ce que les utilisateurs puissent bénéficier de choix de services protégeant mieux les données. Autrement dit, vive le moteur de recherche ! Tel est le sens d'un amendement déposé par notre collègue Claude Raynal, adopté par la commission des lois avec la bienveillance de son président et de sa rapporteur. Sur ces sujets éminemment modernes, le Sénat discute et le Sénat amende ; le Sénat prouve ainsi son utilité au Gouvernement, comme toujours sur la question très importante des

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance de masse en ligne ont précipité la fin du mythe originel de l'Internet, lequel s'est révélé un instrument de puissance échappant à l'Europe,

Mais notons qu'il aura fallu six ans, le sujet ayant fait l'objet d'un intense lobbying transatlantique. Certes, la vision de la diffère entre l'Amérique et l'Europe, mais il y va avant tout d'enjeux de pouvoir et de domination économique. Des lobbyistes contestent les mesures prises par la Commission européenne pour lutter contre les abus de position dominante et les pratiques déloyales des plateformes horizontales dont l'intermédiation est quasi incontournable. Mais les traitements des masses de données et les progrès de l'intelligence artificielle exigent une transparence absolue des plateformes et des algorithmes utilisés, seule condition de la neutralité. De même faut-il garantir une liberté de choix des fournisseurs de logiciels ou de services nécessaires au fonctionnement de ces derniers. S'agissant des marchés publics portant sur le traitement des données de nos administrations, nous exigeons un surcroît de rigueur du Gouvernement dans le choix des prestataires, notamment lorsqu'il s'agit des données publiques dites sensibles.

a bien failli confier l'administration de nos données fiscales à un acteur privé dont les liens avec des agences de renseignement étrangères sont de notoriété publique. Eh oui ! L'Europe doit donc se doter d'un régime très exigeant de protection des données, incluant les conditions de traitement de ces données, mais aussi, demain, les technologies de protection de la confidentialité, qui représentent les nouveaux instruments de la souveraineté pour l'Europe. je ne vois pas de stratégie pour l'internet des objets. Pourtant, les objets connectés envahissent déjà notre quotidien, se développent dans des domaines aussi sensibles que la santé, les transports, l'environnement, l'énergie ; avec eux grandissent les inquiétudes quant aux usages qui peuvent être faits des données recueillies et quant à la sécurité des dispositifs. Il faut donc une régulation pour renforcer cette sécurité et en même temps promouvoir une politique industrielle dynamique dans ce domaine, assortie, d'ailleurs, d'un droit au « silence des puces », c'est-à-dire à la désactivation. la désactivation. La protection et la sécurité des données personnelles devront aussi s'accompagner d'une obligation de localisation et de traitement des données sur le territoire de l'Union. tout dernier mot : préparant aujourd'hui un rapport sur la formation au numérique, je confirme ce qui a été exprimé, plus tôt, à cette tribune, à savoir l'inquiétude des entreprises et des collectivités,

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi ne doit pas seulement être considéré comme la conséquence du règlement européen relatif à la protection et à la libre circulation des données. C'est un texte très important, pas simplement technique, mais- mon collègue Loïc Hervé l'a dit -très politique. en effet de nombreux enjeux contemporains ayant trait au numérique : enjeux juridiques, avec la protection des données personnelles ; enjeux économiques, avec la stimulation et la diffusion de l'innovation enjeux scientifiques, avec la profusion de données rendues accessibles, ce qui ouvre de nouveaux champs d'exploration, notamment pour la recherche publique ; enjeux sécuritaires et géopolitiques, avec l'échange de données entre les États pour des motifs de maintien de l'ordre public ; enjeux

prise. Ce projet de loi tendant à modifier en profondeur la loi fondatrice de 1978, il est en premier lieu légitime de veiller à ce que les droits et libertés inscrits à l'article 1 de cette grande loi soient toujours effectifs. Car le renversement de paradigme qui est opéré, avec le passage d'une logique de déclaration ou d'autorisation préalable à une logique de responsabilisation, mais aussi de contrôle des acteurs mettant en oeuvre des traitements, ne doit bien sûr pas se traduire par un affaiblissement des libertés individuelles et publiques. Le Sénat, Le Sénat, on le sait, a toujours porté une vigilance aiguë au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, droit fondamental désormais inscrit à part entière dans l'ordre juridique européen. Ce fut en particulier le cas lors du débat que nous avons eu sur le projet de loi pour une République numérique. Le groupe socialiste et républicain s'est bien sûr inscrit naturellement dans cette tradition ; c'est pourquoi nous proposons un certain nombre d'amendements sur les algorithmes ou les données sensibles- nous y reviendrons dans la soirée. Indépendamment du développement des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, qui irriguent désormais notre société, il ne faut jamais perdre de vue que la loi de 1978 est intrinsèquement et premièrement une loi protectrice des libertés individuelles et publiques. C'est une « loi socle », équilibrée, riche, reconnue et rassurante, aussi bien pour les acteurs concernés que pour les citoyens. En tant que parlementaires, nous devons nous assurer qu'elle ne soit pas affadie ni dépréciée.

mais aussi des collectivités territoriales, en amont, et la consolidation du volet répressif, en aval : plaintes, contrôles et sanctions. Cette mutation substantielle est directement induite par le changement de paradigme que j'ai précédemment D'ailleurs, la CNIL a d'ores et déjà anticipé ces évolutions, en produisant des instruments de droit souple : les « packs de conformité », la valorisation des démarches, les codes de bonne conduite. Néanmoins, il est évident que l'application du RGPD, combinée à la démultiplication de ses missions, représente vraiment un changement d'échelle pour cette autorité administrative indépendante. Par conséquent, afin que la CNIL puisse mener à bien son action et que, par son intermédiaire, nous continuions à maintenir un haut niveau de protection des données personnelles,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord remercier Mme la sénatrice Joissains, rapporteur

Au contraire, le souci avec lequel ce texte a été préparé- j'y reviendrai -témoigne du profond respect que nous avons pour le Parlement- je tiens ici à le redire.

dans un même texte. Évidemment, tout ceci donne des choses assez complexes, et vous soulignez l'intérêt d'utiliser les marges de manoeuvre, pour traiter notamment la question de l'âge du consentement- là encore, j'avais, me semble-t-il, répondu par anticipation, et nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir. également mention de la charge nouvelle qui pèse sur les collectivités territoriales ; vous souhaitez- je vous cite -un « accompagnement adapté

le sénateur Ravier, je ne partage pas tout à fait les propos que vous avez prononcés. Vous avez bien entendu fait allusion à, aux GAFA,

Au-delà de cette nécessaire prise en compte du problème au niveau européen, notre ambition, dans le cadre de ce texte, est bien de faire respecter nos valeurs telles qu'elles transparaissent dans la loi de 1978. Le rôle que la France a mené dans les négociations européennes a bel et

Madame la sénatrice Carrère, vous avez souligné, autour des notions de défi et de changement de paradigme, l'importance d'un meilleur accompagnement par l'État

à la création de droits de propriété de l'individu sur ses données ; nous ne voulons pas d'une patrimonialisation de celles-ci. Mais le RGPD renforce évidemment les droits des individus sur leurs données.

cette mise à distance au fait que nous n'aurions pas suffisamment répondu aux TPE et aux collectivités territoriales. L'ordonnance que nous proposons n'a rien à voir avec la non-réponse que vous pensez

de souligner le travail qu'ont accompli les services de la Chancellerie dès le mois d'août. Nous ne sommes pas dans l'impréparation que d'aucuns ont bien voulu relever. Dès l'adoption de la loi sur le rétablissement de la confiance, que j'avais eu l'honneur de vous présenter, nous nous sommes immédiatement mis, avec l'ensemble des services de la Chancellerie,

J'y vois précisément l'illustration de l'intérêt d'un cadre européen. Le projet de loi de transposition prévoit justement des mécanismes permettant à la CNIL de prêter son concours aux autres autorités de protection de données

nous avons expressément fait. Nous considérons la loi de 1978 à la fois comme un symbole de la représentation des valeurs portées par la France, mais aussi comme un cadre lisible qui nous semble essentiel. Madame la sénatrice Benbassa,

Un rapport de la Cour des comptes rendu, je crois, en 2016 a montré que la CNIL avait déjà obtenu des moyens importants

la suppression des sanctions et la nécessité que la CNIL porte un regard particulier- nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir -sur ces collectivités territoriales. Monsieur le sénateur Hervé,

Vous avez développé le problème de l'absence de stratégie pour l'Internet des objets, en soulignant l'importance à la fois d'une régulation pour renforcer la sécurité et d'une stratégie pour promouvoir les entreprises innovantes.

un processus assez fort d'accompagnement des élèves aux nouvelles stratégies du numérique et que toute la démarche de responsabilisation des acteurs que nous souhaitons par ailleurs promouvoir doit évidemment être articulée avec la lucidité et la vigilance des citoyens ; c'est un point qui mérite d'être travaillé.

en appelant à une vigilance aiguë quant à la protection de la vie privée des citoyens. C'est, là encore, un point que nous partageons. Je ne sais pas si nous aurons des désaccords au fur et à mesure de l'examen du texte, mais nous nous

Dans, Romain Gary écrivait : « Ce qu'il y a de bête avec la maturité, c'est qu'elle vient toujours trop tard. » Je voudrais faire le pari qu'avec vous, la maturité des quarante ans ne viendra pas trop tard et que nous saurons ensemble travailler pour aller vers plus de progrès et de protection des citoyens ! La discussion

intervertir le débat sur l'article 6 et celui sur l'article 5, en utilisant l'article 44, alinéa 6, de notre règlement,

5 fait référence à ce paragraphe. Imaginez un seul instant que vous adoptiez l'article 5 et que vous rejetiez l'article 6 : qu'adviendrait-il de cette référence à un paragraphe III de l'article 6 qui n'aurait pas été adopté ? C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande instamment de soutenir la demande que je forme en direction de notre président de séance pour que la réserve soit acceptée, à condition, bien entendu, que Mme la ministre